La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, ils ont à créer une garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social, présenté par Monsieur Patrick Kanner, et plusieurs de ses collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 4 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de nos collègues du groupe socialiste vise à réduire le nombre de chômeurs de longue durée en investissant dans les emplois de la filière écologique et le lien social au 4ème trimestres 2021 le nombre de chômeurs était évalué à 2, 2 millions de personnes en France, dont environ 700000 chômeurs sans emploi depuis au moins un an, auxquels il faut ajouter 2 millions de chômeurs sans emploi qui ne rentrent pas dans les critères de Pôle emploi cette proposition s'appuie sur les travaux des associations et, notamment, de l'ONG ATD quart Monde, que je remercie pour son travail et d'ailleurs les recherches, ils ont fait sur le coût du chômage de masse pour la société, il est légitime de s'interroger sur le coût pour la société de maintenir près de 4 millions de personnes sans emploi, le coût pour la société est loin de se limiter à la prise en charge de l'indemnisation chômage, il s'agit aussi d'une perte de création de richesse d'une perte de rentrées de cotisations sociales pour la sécurité sociale, d'une baisse de la consommation et des dommages psychosociaux pour des familles entières, lorsque ma collègue Katia pour Poli a rencontré les anciens salariés de Bridgestone, toujours à la recherche d'une solution elle partage avec eux qu'il ne s'agit pas seulement d'un coût financier mais aussi et surtout d'un coût humain, contrairement au président de la République, qui considère qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, je voudrais rappeler que ce n'est pas aussi simple et dans la vraie vie, la perte d'un emploi, c'est aussi la perte des relations sociales, la perte de mise en pratique de ces talents, la proposition de loi apporte un discours positif, au lieu de culpabilisation des chômeurs, en permettant à chaque personne au chômage depuis plus d'un an de bénéficier d'un emploi dans le secteur social et celui de la reconstruction écologique, le texte propose une refonte de la fiscalité avec le rétablissement des impôts de production, l'instauration d'un impôt de solidarité sur la fortune, sous la forme d'un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, la suppression de la flat tax et l'augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières, une série de mesures, mes chers collègues, que nous soutenons, pour les avoir défendus à chaque discussion budgétaire mais nous ne pouvons que regretter que cette réforme de justice sociale n'ait été entreprise entre 2012 et 2017 face aux défis des nouvelles technologies de la révolution informationnelle, il est indispensable pour nous de proposer des perspectives durables avec un accompagnement, une formation des privés d'emploi face à la précarité de l'emploi, il est nécessaire d'apporter des solutions qui ne se limite pas au recrutement de 200000 CDD c'est le sens de notre proposition de sécurité de l'emploi et de la formation associée à un plan de recrutement publiques et une augmentation générale des salaires de 30 % dans la fonction publique à l'augmentation du SMIC à 1500 euros il faut également accorder des droits nouveaux dans les entreprises pour les salariés et pour ces raisons, il faut abroger un certain nombre de lois notamment les loi El Khomri les ordonnances Macron et revenir sur la réforme de l'assurance chômage, nous regrettons donc que cette proposition de loi n'aille pas suffisamment loin, nous l'avons dit d'ailleurs, en commission, c'est pour toutes ces raisons qu'au niveau du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, nous nous abstiendrons sur cette PPL je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Brigitte Devésa pour le groupe Union centriste pour 6 minutes

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente des affaires de la commission sur les affaires de la commission sociale, mes chers collègues permettez-moi de saluer la clarté du rapport de monsieur Jean-Luc Fichet, ainsi que le groupe socialiste, écologiste et républicain pour avoir inscrit cette proposition de loi visant à créer une garantie d'emploi pour les chômeurs de longue durée, dont les activités utiles à la Russe construction écologique et au développement du lien social. Une proposition de loi qui a certes le mérite de proposer un projet de société, de s'engager pour la lutte contre le chômage, d'y apporter des réponses et de permettre de rappeler dans cet hémicycle, que le chômage de masse sur plusieurs générations, mine la société de l'Intérieur et qu'à force de s'inscrire dans le paysage français, il a fini par rendre l'élite du pays apathiques décourager, voire pire, à s'habituer au chômage de masse et à se réjouir d'un taux à 8 %. Le plan de lutte contre le chômage de longue durée, décliné dans cette proposition de loi de manière exhaustive détaillée financièrement avec une précision et un sens de l'équilibre qui fait de ce texte, une proposition de loi aux allures de projets de loi, voire peut-être même un programme présidentiel, la commission des finances aurait d'ailleurs pu être sollicité alors vouloir garantir aux chômeurs de longue durée un emploi est une attention louable, comment s'y opposer, d'autant que l'emploi serait en droit constitutionnel jeudi serait parce que bon nombre de juristes estiment qu'il y a eu à la Libération, une confusion entre les termes droit l'emploi et droit au travail, autre attention louable, celle de trouver de la main d'oeuvre et là où il en manque et l'on sait que les besoins sont nombreux d'ici 2030 d'après l'Insee, la moitié des agriculteurs en activité vont partir à la retraite. Dans le secteur des transports routiers, on compte entre 40000 et 50000 emplois non pourvus les besoins pourrait atteindre les 100000 postes dans les 5 ans à venir. Quant aux armateurs et nous alerte : qu'est ce qu'il dit, ces armateurs, bien que les officiers et les marins manque sur ce point, la portée de votre dispositif ne semble pas apporter trop de solutions. Selon un rapport de la Direction des statistiques et de la recherche, la Darès en 2020 parmi les 30 métiers les plus en tension dans le marché du travail, on compte les ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les charpentiers, les couvreurs, les plombiers, les métallier les chaudronniers, permettez-moi de dire la proposition de loi qui nous est présenté, mes chers collègues, viendra-t-elle pouvoir ses métiers et ces secteurs en manque, c'est des questions, le métier de couvreurs est-il alors considéré comme une activité utile à la reconstruction écologique si l'entreprise n'est pas qualifié ou ne se spécialise pas dans leur ouvrage par exemple du toit à la chaux. Par conséquent, voici la principale opposition à cette PPL. Vous élaboré un plan financier complexe par l'instauration donna notamment d'un nouvel impôt, dit de solidarité sociale et climatique sur le capital. Pourquoi pas vous accélérez des expérimentations sur le terrain, modifiant la nature et le rythme de celles-ci. Mais vous à Lourdes il c'est aussi le budget de l'État de 7 milliards d'euros pour la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et l'abaissement de la contribution économique territoriale pour financer vers une autre aura rien tation pardon vers les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social, orientation certes louable mais arbitraire, certains diront idéologique ce qu'Europe peine le rapport de monsieur Jean-Luc Fichet lorsqu'il estime que certaines entreprises pourraient être exclus de la liste des entreprises socialement et écologiquement responsable alors qu'elles opèrent dans des secteurs tout de même stratégique, vous en conviendrez, pour l'économie française ou sont créatrices d'emplois ou de forte valeur ajoutée. Par cette proposition de loi, vous avez voulu introduire une hiérarchie des activités entre secteurs essentiels et non essentiels, ils sont ainsi la protection de l'environnement et les métiers du lien social devant toute autre activité. D'ailleurs, il y a un flou sur la définition de ce que vous appelez activités utiles à la reconstruction écologique ou activités utiles au développement du lien social. Je me demande seulement si le secteur des cafetiers et restaurateurs et compris dans des activités utiles au développement du lien social, parce que si cela n'est pas le cas, alors comme à Narbonne, souvenez-vous, les restaurateurs devront prendre de leur propre initiative, l'augmentation de 30 % des salaires pour attirer la main-d'oeuvre la préserver et faire face aux pénuries. Cette hiérarchisation et contestable. On pourrait alors proposer une PPL garantissant un emploi aux chômeurs de longue durée pour des activités utiles à la culture à l'éducation, développement du sens civique et citoyen par exemple. Quoi qu'il en soit, une autre question se pose : comment pouvons nous présenter un texte visant à orienter sur les métiers de demain, comme la reconstruction écologique sans évoquer une seule fois la question de la formation, vous avez préféré recourir à la création de nous à l'impôt, impôt qui, comme votre PPL d'ailleurs doit être acceptable parce qu'elle contient dans son intitulé Les mots solidarité sociale et climat, il est vrai que les expérimentations les dispositifs existants comme l'insertion par l'activité économique ou les contrats aidés peuvent être améliorées et que les périmètre stations peuvent toujours faire l'objet de réflexions, mais vous me permettrez, mes chers collègues, de ne pas entrer plus en détail dans les mesures financières de cette proposition de loi quand le groupe Union centriste que je représente, aujourd'hui, n'en partage pas la philosophie, la philosophie générale, c'est pourquoi, chers collègues, notre groupe ne votera pas favorablement ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente, mes chers collègues, l'année 2021 a connu une baisse importante du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a ainsi reculé de 12,6 % ce qui représente 480000 personnes au moins, il semblerait également que le chômage de longue durée, après avoir atteint un pic au 1er trimestre 2021 est entamé une légère décrue en fin d'année, il représente toutefois encore 49,6 % du total des demandeurs d'emploi, par ailleurs, si l'on regarde les chiffres de plus près, le nombre de chômeurs inscrits depuis au moins 2 ans, à augmenter les personnes les plus éloignées de l'emploi sont les premières frappés par les crises et souvent les dernières à bénéficier de la reprise, mais derrière ces chiffres égrenés régulièrement nous n'oublions pas qu'il y a des personnes détruite par des carrières brisées, des fractures de vie qui ont perdu confiance en elles et parfois leur dignité, nous connaissons les conséquences humaines et sanitaires de l'absence d'emploi de plus en plus d'associations, d'organisations syndicales et de professionnels de santé nous alerte sur le traumatisme que constitue le chômage et ses effets délétères sur la santé physique et psychique, comme le rappelait un avis du CESE en France où la population se distingue par un véritable investissement dans la valeur travail qui vient parfois supplanté d'autres dimensions de la vie, perdre son emploi c'est perdre son identité sociale voir sa valeur sociale, coupable d'avoir perdu leur emploi, ces personnes à terme s'isolent socialement le traumatisme du chômage se traduit également par une surmortalité par une détérioration de la santé physique et mentale et par des conduites addictives, plus fréquente quand ils durent plusieurs années, le chômage fait naître chez beaucoup un sentiment d'exclusion, un traumatisme que les psychiatres assimile à une période de deuil dans ces conditions, nul doute que la lutte contre le chômage de longue durée doit être une priorité, c'est l'objet de la proposition de loi présentée par le groupe socialiste, écologiste et républicain qui vise à mobiliser plusieurs dispositifs d'insertion professionnelle nous souscrivons pleinement à l'objectif poursuivi par nos collègues, personne ne doit, ne doit en effet s'accommoder d'un taux de chômage récurrent pour autant penser ce combat sous le seul prisme des emplois aidés, risque de nous faire passer à côté de l'enjeu majeur que notre pays pays doit relever les emplois aidés sont malheureusement bien souvent des contrats précaires et constitue malheureusement aussi une aubaine pour certains employeurs dans le secteur marchand, seuls 25 % des contrats aidés débouchent ensuite sur un emploi, nous regrettons également que la proposition de loi ne comportent pas de volet formation piliers pourtant indispensables le 1er ministre a annoncé en septembre dernier, sa volonté de former un virgule 4 millions de demandeurs d'emploi en 2022, et pour éviter que la reprise ne laisse au port au bord de la route, les publics vulnérables l'emploi devrait déployer le parcours demain de remobilisation expérimenté depuis quelques mois, pour permettre aux chômeurs sans activité depuis 2 ans ou plus, de retrouver un emploi ou une formation dans une période de 6 mois, s'agissant enfin de la pérennisation du dispositif territoires zéro, chômeur de longue durée qui est proposée, elle risque d'être prématuré, d'autant que la loi du 14 décembre 2020 a prévu une évaluation de l'expérimentation, afin qu'elle puisse être prolongé et élargi ou pérenniser toutes ces raisons, le groupe RDSE s'abstiendra majoritairement sur cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Monique Lubin, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame

madame la présidente de commission monsieur nouveau sur le rapporteur. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Alain Supiot dans l'un de ses articles, dénonçait le renforce le renversement qui consiste à traiter le travail non pas comme la cause mais comme un effet de la richesse avec la proposition de loi que nous présentons aujourd'hui le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat s'oppose à ce renversement, nous rappelons que le travail est cause de richesses, il est avant tout parce qu'il permet de produire directement en termes de biens et de services en ce sens c'est un bienfait dispensés par le travailleur s'en est également un parce que toute personne qui travaille et qui, pour ce faire, bénéficient d'un droit dédié et protecteur est en mesure de contribuer à la vie de la société et à la qualité du tissu social, dans les meilleures conditions, à contrario, le chômage de masse est à plusieurs titres au profondément délétère, il a d'abord des coûts psychosociaux et en terme de santé publique, il est et les finances publiques, affaiblissant les recettes de l'assurance sociale et nécessitant par exemple la mise en place de politiques d'accompagnement, même dans des périodes comme celle que nous traversons, où les chiffres de l'emploi sont meilleures, et je dirais peut-être surtout dans des périodes comme celle-ci, nous nous devons d'être vigilant et d'impulser des politiques exigeante au profit des personnes encore enlisées dans le chômage de longue durée, derrière ces données sympathique se cache en effet certaines vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, nous constatons en effet une amélioration de la situation de l'emploi, mais il y a encore 5 millions 600 1000 personnes inscrites au chômage, concernant par exemple les radiations, elle contribue à la statistique optimiste mise en avant par le gouvernement, puisqu'elle représente 9 4 sorties des des des listes de Pôle Pôle emploi or, leur nombre a bondi de 45 % depuis un an, posons-nous la question du rôle que joue la réforme de l'assurance chômage dans cet accroissement, nous avons un devoir de volontarisme pour ce qui alimente encore les chiffres du chômage et ceux qui sont sortis des radars, il n'y a pas de personnes inemployables, mais des compétences mal identifié et mal valorisé la présente proposition de loi proposée par notre président du groupe, Patrick Kanner a donc pour objectif de contribuer à lutter contre ce phénomène et de créer une garantie à l'emploi pour les personnes qui en ont été privés durablement nous partons en effet d'un constat : le besoin travail est inépuisable, mais les travailleurs se heurtait à une structuration du marché du travail défaillantes, je me permet d'ailleurs de rappeler ici que non les entreprises ne pâtissent pas massivement d'une situation dans laquelle les postes seraient non pourvus, ni d'une pénurie de main d'oeuvre, Pôle emploi a en effet publié le 10 février dernier une étude soulignant qu'en 2021 sur les 3 1000000 1000000 100 offres d'emplois qui étaient déposées et clôturées, seuls 6 % des recrutements se sont soldées par l'abandon du recrutement, faute de candidats, selon le préambule de la Constitution de 46, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, c'est pour y tendre que nous présentons la présente proposition de loi pour ce faire, nous nous appuyons sur 3 piliers : la montée en puissance de l'expérimentation territoire zéro, chômeur de longue durée, le développement de l'insertion par l'activité économique, le développement des contrats aidés, on ne présente plus, ces dispositifs expérimentation, le choix est cependant trop souvent fait en France dans le cadre des politiques publiques de ne pas les consolider, ni les conforter une fois installé, et ayant fait leurs preuves, au contraire, les pouvoirs publics choisissent plutôt l'option de passer à l'expérimentation ou au dispositif suivant, il faut aller plus loin avec territoires zéro, chômeur de longue durée et l'insertion par l'activité économique, notamment, nous avons par exemple des éléments d'une politique à destination des chômeurs de longue durée sur lesquelles il faut faire fond il comporte en effet une dimension formation les plus précieuses, qu'elle soit formalisé en tant que telle qu'elle est une dimension expérience par ailleurs si un amendement bienvenue du rapporteur attends tend à remplacer la conditionnalité verte pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi par une approche essentiellement incitative, il n'en reste pas moins que la présente proposition témoigne de notre souci de la protection de l'environnement, c'est à cela que nous devons tendre, il en va de même pour le 3ème amendement du rapporteur qui concernant les contrats initiative emploi réserve la conditionnalité de neutralité carbone aux entreprises de plus de 250 salariés dans le cadre du développement de l'économie sociale et solidaire que nous soutenons en nous inscrivant soutien au travail du tissu associatif, des coopératives et de toutes les entreprises concernées, nous prenons en effet le verdissement de tous les emplois susceptibles de connaître une telle évolution, notre approche est bien une approche systémique et c'est pour cela qu'elle repose sur 3 piliers différent, c'est également la raison pour laquelle nous reprenons avec plaisir l'observation qui nous a été faite en commission selon laquelle notre proposition de loi relèverait également du texte de politique générale, avec un volet de politique sociale et un volet de politique fiscale, c'est très exactement cela face à l'ampleur des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter de politiques de courte vue et sans ambition, l'intérêt de notre démarche et par ailleurs de s'appuyer sur des expérimentations et des manières de procéder nécessitant sur le temps, un travail sur le temps long, impliquant les acteurs locaux qui ont pris le temps de bien connaître leur territoire et de développer une vision le concernant ces acteurs ne sont pas uniquement investi dans une démarche volontariste, ils doivent également faire démonstration de l'existence d'un projet pour le territoire et les populations concernées, nous affirmons en effet au diapason du secteur associatif et des parties prenantes que loin des logiques descendante, c'est bien par la co-construction penser et menée au niveau local avec des modalités partout différentes que nous sommes susceptibles de trouver les moyens de faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui et je terminerai en remercions bien évidemment notre rapporteur et notre président de groupe pour le travail fourni sur cette proposition de loi. Mais si sa collègue, la parole est à monsieur Martin lévrier. Pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes indépendants pour 4 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre pays connaît un problème structurel de chômage de longue durée depuis 40 ans. En 2020, selon l'OCDE, les chômeurs de longue durée, représenté 36,7 % des demandeurs d'emploi en France, un taux en chute de 8 points depuis 2017 preuve une politique de l'insertion efficace et volontaire pour autant, et bien que la reprise économique se confirme, beaucoup d'entreprises peinent à recruter dans le donc dans de nombreux secteurs, souvent en manque de main-d'oeuvre, avant la crise, comme vous, Monsieur le Président Kanner, j'affirme qu'il n'y a ni fatalité au chômage ni impuissance de politiques économiques, c'est en ce sens que vous avez déposé la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, celle-ci, composée de 8 articles vise à garantir des emplois pour les chômeurs de longue durée dans les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social de notre pays, ce texte l'exploration, l'expérimentation territoire zéro, chômeur de longue durée, définirait un objectif de 100000 contrats supplémentaires relevant de l'insertion par l'activité économique d'ici à 2023 instituerait 200000 emplois aidés CUI, CAE ciblée sur les éco-activités. Pour financer ce texte il consacrerait l'annulation de la baisse de 10 milliards des impôts de production, acteurs et la mise en place d'un impôt solidarité sociale et climatique sur le capital supprimerait le prélèvement forfaitaire unique, introduit en 2018 acteurs et la mise en page, le dit : pas de forfait, le taux de la taxe des transactions financières, je me dois-je rappeler ici que la forte baisse du chômage est en partie liée à la visibilité fiscale retrouvés par les entreprises, ces 5 dernières années, non, le chômage n'est pas une fatalité, preuve en est, puisque notre majorité, a contribué à la baisse du taux du chômage lui permettant d'atteindre les 7,4 % au 4ème trimestre 2021, son plus bas niveau depuis 2008 et ce n'est pas tout : Emmanuel Macron, a fait de l'insertion par le travail, un des piliers de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, une volonté définie dans le pacte d'ambition pour l'y a eux donc un des objectifs était d'augmenter de 25 %, le nombre de postes dans ce secteur d'ici à 2022 offrant une opportunité à 100000 salariés supplémentaires. Et c'est pour répondre aux tensions de recrutement que le gouvernement a lancé il y a 5 mois, un plan ambitieux de 1,4 milliards d'euros avec un volet inédit dédié à la formation de ce public dans une logique d'aller vers Pôle emploi ainsi recontacter tous les chômeurs de longue durée, fin 2021 et les packs de remobilisation seront déployés partout d'ici juin, de plus, le plan prévoit également de mobiliser 240 millions pour étendre les aides à l'embauche de 8000 euros, dans le cadre des contrats de professionnalisation, aujourd'hui réservée aux jeunes 100000 d'entre eux ont ainsi retrouvé un emploi, entre octobre et novembre ont mis 2021 les dispositifs en vigueur sont efficaces, l'expérimentation territoire zéro chômeur a elle aussi prouvé son efficacité aussi, nous avons déjà voté dans cette assemblée, son renforcement, souvenez-vous, c'était il y a un an, la loi de décembre 2020 a élargi le dispositif à 50 nouveaux territoires, en plus des 10 initiaux, la durée de l'expérimentation a été étendue à 5 ans et son financement est assuré par les fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, dont le rôle était tendue également. Parce que les dispositifs mis en place par le gouvernement répondent déjà aux objectifs de ce texte et que nous sommes en désaccord avec le financement que vous proposez, parce que le coût de celui-ci n'est pas soutenable et que nous avons prouvé qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec moins, notre groupe votera contre cette PPL je vous remercie.

minutes. La présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, les chiffres du chômage sont au plus bas depuis 15 ans fin 2021, la population active, comptait 7,4 % de chômeurs, chiffre légèrement supérieur à la moyenne de la zone Euro, situé à 7 la dynamique actuellement observé des un schéma favorable pour parvenir, la proposition de loi que nous examinons propose de lutter contre le chômage de longue durée en instaurant une garantie d'emploi grâce à des centaines de milliers d'emplois subventionnés par l'État et financé par une réforme fiscale consistant à rétablir l'ISF et annulé l'allégement de 10 milliards d'euros des impôts de production des moyens qui apparaissant en réel décalage avec la situation actuelle, nous savons que le chômage touche principalement les moins diplômés, les moins qualifiés, les personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes de santé, les jeunes et les seniors, nous savons également que les difficultés d'accès au logement et à la mobilité sont parfois des freins qui elle voit une et demandeurs dans l'emploi du marché du travail, nous sommes enfin que le nombre de chefs d'entreprises connaissent, qui connaissent des problèmes de recrutement est important, nous pouvons réduire les distorsions entre marché de travail et compétences des demandeurs de d'emploi avec la formation et l'accompagnement vers l'insertion, formation des jeunes avec l'apprentissage dont nous connaissons les excellents résultats mais également avec les nouvelles mesures lancées par le gouvernement, le contrat d'engagement jeune qui s'inscrit dans la côte unité du plan, un jeune une solution mise en place en juillet 2020, qu'il faudra bien sûr évaluer, il apparaît également essentiel de renforcer le taux d'encadrement des demandeurs d'emploi par des conseillers du service public de l'emploi, la création de 1000 400 nouveaux postes en 2022 va dans ce sens mais nous devons aller plus loin, il existe de fortes disparités entre les territoires, certaines agences compte un conseiller pour 350 demandeurs d'emploi, si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté, il faudrait augmenter ce taux de moitié, nous devons également renforcer la concertation avec les partenaires sociaux, proposer des solutions personnalisées aux problèmes de logement, problème de santé de mobilité, de maîtrise de la langue française et parfois d'addiction, une constellation de dispositif de soutien existe, il serait utile de réaliser une carte que biographie de ces aides de l'État et des collectivités, il faudrait évaluer leur efficacité et leurs modalités d'attribution et des reprises d'activité qu'ont trouvé du travail peut se révéler coûteux en terme de frais de transport, de garde d'enfants ou de déménagement, il est indispensable de lever ces obstacles par une insertion durable dans l'emploi, je ne suis pas contre le dispositif territoires zéro, chômeur de longue durée, loin de là, mais l'assurance de sa neutralité économique est un préalable à sa généralisation, je ne pense pas que le chemin du plein emploi passe par une un un mot un amoncellement de dispositifs coûteux et lisible, mais par une meilleure coordination entre le politique de l'emploi et le marché du travail, redonnons du sens et de la valeur au service public de l'emploi en améliorant la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et puis profitons de l'expérience des seniors, un atout précieux pour de nombreux chômeurs de longue durée, le développement du mentorat à tous les âges de la vie est un facteur de lien social et de réussite collective ne le négligeons pas le groupe, les indépendants républiques et territoires ne partage pas le projet de société, porté par cette proposition de loi ni dans sa dimension sociale, mais dans sa dimension fiscale. Merci de votre attention, merci. La parole est à Madame, Frédérique Puissat pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la présidente de la commission d'affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie le président Patrick Kanner et ses collègues d'avoir mis à l'ordre du jour de ce soir sa proposition de loi visant à créer une garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement, il y a social. Notre collègue Jean-Luc Fichet a conduit plusieurs auditions et le jour, je le remercie de son travail au-delà de nos divergences sur lequel je reviendrai bien entendu ce texte mis en exergue la valeur travail pour l'importance transcende nos groupes politiques et les rangs de cette assemblée, le travail est facteur de progrès social, il est l'axe de lutte contre les inégalités, perdre un emploi entraîne une altération du nouveau devis et demeure un traumatisme social et quand la perte d'emploi, dur et que les mois s'installe, les motivations s'affaiblisse pour laisser place à un certain désespoir qui peut s'avérer être un obstacle supplémentaire au moment de postuler à des entretiens d'embauche notamment au-delà de ce point de convergence, les points de divergences existent et ils sont forcément nombre d'abord sur le fond. Je suis un peu surpris si vous voulez annoncer mon cher collègue, rapporteur de l'article 1er de cette proposition de loi qui pérennise le dispositif territoires zéro chômeur longue durée alors même que l'encre du projet de loi visant à prolonger son expérimentation est et à étend le dispositif est à peine sèche, autre proposition permet donc de rappeler la proposition de loi de 2020 votée par une très grande majorité de cet hémicycle dans les sorties, IV, V et VI concernés le dispositif territoire zéro chômeur et qui rappelaient que ce dispositif avait à sa création en 2016 3 objectifs : le 1er éradiquer le chômage de longue durée dans les 10 premiers territoires expérimentaux, le 2ème mesuré les effets positifs du retour à l'emploi, le 3ème vérifier l'équation financière sur lequel il repose les coûts Directs et indirects de la privation durable d'emplois ne sont pas supérieurs au coût d'un emploi rémunéré au SMIC, vous le savez, je me permets, mes chers collègues d'insister parce que j'entends dans cet hémicycle depuis un certain temps que ce dispositif a effectué un certain nombre de réussite je me permettant d'assister pour vous dire que les évaluations de ce dispositif sont nombreuses sont coûteuses, monsieur le Ministre, quasiment 100000 euros, donc on n'a pas lésiné effectivement sur ces évaluations, mais elles sont contrastées, si elle n'avait pas été contrastées, nous aurions bien entendu inscrite définitivement ce dispositif dans dans la réalité de notre paysage social comme elles sont contrastées : nous avons fait le choix volontairement et ensembles de prolonger cette expérimentation et de l'étendre à un certain nombre de dispositifs, alors j'ai bien vu, chers collègues, que vous aviez nuancer votre 1er texte en énonçant le fait que vous souhaitiez aller au-delà des 60, territoire, enfin en tout cas des 50 plus 10 avec effectivement à cliquer que vous souhaiteriez levé puisque je vous rappelle quand même que la ministre s'était engagé en CMP, à ce qu'il n'y a pas de limite, sur les 60 territoires et qu'on puisse étudier au cas par cas, la situation vous avez levé le de créer, c'est-à-dire que vous n'avez pas poussé la refonte de l'expérimentation, contrairement à ce qui ce qui s'était passé préalablement mais en tout état de cause, nous considérons que ce dispositif doit encore faire ses preuves et c'est pour ça que nous l'avons prolongé l'article 2 et 3 de ce texte, vivez rapidement vise à augmenter les dispositifs et des plus 100000 postes en acier, eux, d'une part, et plus 200000 emplois c'est ici à eux en collectivité ciblée sur des emplois des collectivités, nous partageons le fait que le dispositif d'accès et retour employes sont fondamentaux, notamment nous appuyons sur les structures de service public de l'emploi et les outils d'insertion professionnelle, mais de là, a décrété que le besoin des demandeurs d'emploi nécessite de quasiment doubler l'existence des places en SIAE et de doubler les employes, on parcourt ampleur qu'on emploie, compétence, c'est d'une part nié les forces humaines disponibles sur le terrain, c'est, d'autre part, ne pas s'attaquer à la racine des problèmes et nos collègues Brigitte Devésa et Maryse Carrère ont souligné, entre autres, les enjeux de formation et c'est enfin, il y a eu ni la réalité des tensions de recrutement en activité classique que nous rencontrons dans nos nombreux secteurs secteurs aujourd'hui quant au second titre de ce texte, nous retrouverons sans surprise des sujets de divergence classique dont une nouvelle forme d'imposition la peau annuelle de solidarité sociale et climatique, la suppression de la flat tax, l'annulation de la baisse des impôts, de production, une hausse de la taxe sur les transactions financières dans la perspective de financer les 17 milliards d'euros d'une mesure pour le moins et malgré tout le respect que nous avons, pour vous, chers collègues, ce sont des divergences d'approche que nous avons et sur lequel nous ne nous retrouvons pas sur la forme, je me permets simplement parce que je l'ai évoqué en commission d'évoquer le tweet de Laurent Grandguillaume à qui le devance ce texte sur l'expérimentation, qui a été très surprise de ce texte de loi quand il est arrivé, je pense qu'il manquait un brin de concertation qui je crois est arrivée après en tout état de cause, pour toutes ces raisons font et forme nous confirmant la position que nous avons eus en commission sociale et nous vous proposerons donc un vote, un vote qui ne sera pas un vote favorable pour ce texte de. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Raymonde Poncet Mons. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le groupe écologiste se félicite que cette proposition de loi du groupe socialiste, nous permettent de débattre d'une approche alternative quant à la lutte contre le chômage, notamment de longue durée, une approche qui prouve que non, on n'a pas tout essayé dans cette lutte, en effet, le principe de la garantie d'emploi et une une des pièces maîtresses d'un cadre théorique élaboré par les économistes de la théorie moderne de la monnaie aux États-Unis, plus spécifiquement par la chercheuse pas l'Nova. Qui rompt avec la théorie néo-classique du taux de chômage d'équilibre de long terme cher à la Commission européenne qui le situe encore à 8 pour 8 2 % pour la France en deçà de ce taux, les salaires réels augmentent rétro et provoquerait inflation et baisse des profits, il faut donc se résoudre à ce taux de chômage ou le faire baisser par des réformes structurelles qui affaiblissent le rapport de force au détriment des salariés assis alors n'est-il de la réforme de l'assurance chômage, une autre façon de faire baisser ce taux réside dans les cadeaux fiscaux en subventionnant les employes et qui ne soutiennent surtout que les profits et les distributions de dividendes assis les exonérations en direction des entreprises se sont révélées hautement inefficace en matière de création d'emplois, à peine 160000 emplois créés, selon le comité de suivi du CICE en 2018, pour un coût cette année-là de plus de 40 milliards, soit une somme bien plus exorbitants que le dispositif présenté ici évalué à 17 milliards en proposant à 5 personnes au chômage depuis plus d'un an, qui ont fait la demande du 9 d'emploi effective à temps choisis payés à minima au SMIC horaire et ceci donc à grande échelle en mobilisant tous les schémas possibles de l'insertion, la proposition de loi rompt avec une pensée économique incapable de juguler le chômage et pose le 1er jalon d'une nouvelle conquête sociale la garantie à l'emploi pour tous les Français, et ce à partir du postulat que personne n'est inemployable nonobstant un accompagnement et une formation et dans le cadre prioritaire d'activité sur les territoires, visant à prendre soin de l'environnement et des personnes et répondant donc à des besoins locaux non satisfait de la transition écologique très intensive en emploi. Des employes porteurs de sens à contrario des boules sites jobs conceptualisé par l'anthropologue David Treiber en effet si la proposition de loi marque une volonté politique rompant. Avec la doxa néo-libérale l'ambition et la mise en oeuvre et bien localiste et par des territoires via une gouvernance partagée, à l'instar effectivement des projets Territoires zéro chômeur dont l'extension à tous les territoires près sera favorisé mais sans exclusive d'autres projets ayant leurs propres spécificités et respectant le code de la garantie d'emploi complémentaire du revenu minimum garanti, la garantie d'emploi pour tout se décline d'abord par l'urgence de mettre fin au chômage de longue durée, drame social absolu principales entrées de la grande pauvreté, de l'exclusion sociale et dont le coût est alarmant, selon l'INSERM, serait responsable de la mort de près de 10000 à 14000 personnes par an en France, il favorise les addictions double le risque de suicide depuis il s'accompagne d'une perte massive de compétences des chômeurs sans même évoquer son impact sur les finances y a plusieurs déterminants sociaux dont le handicap, il représente la un gâchis humain et mine la cohésion sociale, comme le potentiel de croissance des économies, d'après une recommandation du Conseil de l'Union européenne, ce public sera donc la première près priorité de cette garantie parce que la garantie d'emploi incarne une société où l'emploi n'est plus conditionnée aux seuls besoins de rentabilité du capital mais par des besoins communs démocratiquement définies, parce que cette garantie permet la participation de

madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, depuis 1983 le taux de chômage en France n'est jamais passé en dessous de la barre de 7 % même en période de croissance soutenue depuis cette époque, les gouvernements successifs semblent avoir abandonné l'idée que leur action pourrait ramener le pays au plein emploi, on se souvient de cette phrase du président François Mitterrand cinglante aveu de l'échec restées célèbres dans la lutte contre le chômage on a tout essayé. Nous partageons les préoccupations des auteurs de la proposition de loi disant a créé une garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social, il est en effet inquiétant de voir notre société s'habituer à un chômage endémique qui mine la compétitivité économique et la cohésion sociale, toutefois, le texte que nous examinons ce soir est une nouvelle illustration de la capacité des socialistes a abordé le problème du chômage à l'envers. Il s'est installé depuis longtemps un taux de chômage structurel en réalité indépendant des fluctuations de l'activité économique ou même des interventions conjoncturel de l'État, l'argument selon lequel le chômage qu'il soit de longue durée ou pas, or et pour cause, l'absence de garanties à l'emploi et donc le résultat d'une conception qui n'a jamais appris des erreurs commises depuis 40 ans. La France accumule des politiques de l'emploi, basé sur la dépense publique, sans aborder les causes profondes du chômage structurel, cette proposition de loi s'inscrit, hélas dans cette lignée, cette dernière se base sur une interprétation très particulière du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel chacun a le droit d'obtenir un emploi et en conclut qu'il faudrait rendre effective la garantie de l'emploi pour tous, pour tous or le droit d'obtenir un emploi ne s'entend pas comme une obligation de résultat et comme une obligation de moyens, des pouvoirs publics. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelle qu'il appartient au législateur de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés, le travail ne se décrète pas, à moins de sociabiliser toute l'économie privée il n'existera jamais, de garantir l'emploi ce texte présuppose également que la dépense publique serait encore le meilleur moyen de remédier au chômage de longue durée, les articles 3 et 4 réactive ainsi 2000 emplois aidés, c'est une c'est à eux dans le secteur non marchand et réserve les CES, CIE aux emplois qualifiés de verts du secteur marchand, ils ne prennent absolument pas en compte le bilan désastreux. Qui a été fait des emplois aidés par la Cour des comptes en 2018. Abandonnés dans tous les pays comparables à la France, il représente le coup le plus onéreux de toutes les politiques de l'emploi, alors même qu'ils sont inefficaces pour les reins réinsertion professionnelle. En 2020, 37 % des et des personnes, pardon sans emploi peuvent être considérés comme des chômeurs de longue durée. C'est autant qu'en Allemagne, moins qu'en Italie, mais plus que les 32 % en Espagne 24 % Pays-Bas 20 % au Royaume-Uni, sans parler des États-Unis et du Canada, avec seulement 5 si l'on observe le poids de l'État dans chacun de ces pays, il est très difficile de constater un lien entre chômage de longue durée et forte intervention publique, par ailleurs, le groupe socialiste profite de bonnes intentions écologiques et sociales pour promouvoir son idéologie fiscale, ce qui nous apparaît inacceptable les 17 milliards utilisés pour financer ce projet ne feront qu'affaiblir nos entreprises et le Patrimoine des Français : augmenter les impôts de production créer un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en plus de l'impôt sur la fortune immobilière et supprimer le prélèvement forfaitaire unique sur les capitaux mobiliers, voilà des mesures plus guidé par un socialisme fiscal que par une vraie volonté de réduire le chômage, enfin, s'agissant du dispositif territoires zéro, chômeur de longue durée, il paraît plus sage d'attendre la fin d'expérimentation dans 2 ans, plutôt que de le pérenniser, dès maintenant, pour conclure, la fin du chômage de longue durée ne sera pas une réalité en orientant une partie des chômeurs vers des emplois déconnecté de l'économie réelle qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins, précaires, mal rémunérés et financés in fine et par des hausses d'impôts, au contraire, il sera le fruit de réformes structurelles de fonctionnement global de l'économie, prélèvements et transferts sociaux simplification administrative négociations du temps de travail dans les entreprises et surtout politique, de l'éducation et de la formation professionnelle, c'est ainsi que l'on créera des emplois durables dans l'industrie ou la logistique, par exemple, adapté à l'économie aux besoins des Français pour toutes ces raisons, le groupe républicain n'est pas favorable à cette proposition de loi dispendieuses qui ne répond pas aux besoins des personnes sans emploi, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. du débat ce soir, peut-être en écoutant les, les, les intervenants redire un mot sur le fond, parce que ce qui nous réunit, ce soir, c'est la volonté proposer un emploi à tous ces demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 24 mois au chômage, j'ai parlé dans mon propos liminaire, même le président de ce qu'on faisait en matière de Pâques de remobilisation et plusieurs d'entre vous l'ont aussi mentionné, rappelant que le un milliard 4 qui était dédiée par le gouvernement à ce pacte de remobilisation destinée aux chômeurs de très longue durée était en train de porter ses fruits, je, je le dis parce que c'est, c'est sur le fond, le même public que celui qui est visé par la proposition de loi portée par le rapporteur et nous voyons bien que cela fonctionne dans ce qui est fait aujourd'hui tout à l'heure, Martin lévrier, disait-on, on peut sans doute faire mieux pour moins cher, je dirais que au au travers de ce milliard 4 que nous avons mis pour permettre à Pôle Emploi, on a plus de 170 agences pour l'emploi qui aujourd'hui sont déjà en en train de déployer ce pacte de remobilisation toutes les agences le feront d'ici la fin du mois de mai, et bien nous avons, c'est 800000 demandeurs d'emplois de très longue durée, qui seront tous concernés par ce pacte de remobilisation j'étais moi-même à Argenteuil, à Rouen, pour participer à ces séquences de formation où ces demandeurs d'emploi se retrouvent en petits groupes, avec un conseil en évolution professionnelle un conseiller, entreprise de Pôle emploi mais également un psychologue du travail parce que ce que nous savons tous, d'ailleurs, c'est que la situation du demandeur d'emploi, de très longue durée, c'est une situation où il est temps, souvent en difficulté donc l'expression de son besoin l'expression de sa confiance en lui, il a besoin qu'on l'aide à reconstruire tout cela et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec ce dispositif, et je crois Madame le président, si vous permettez, voilà que les éléments et d'ailleurs je je veux en même temps, témoigner, pourquoi je je crois que la position que j'ai entendu de la part de beaucoup de sénateurs et sénatrices qui est de dire, mais sur le fond, cette proposition de loi, les objectifs qu'on peut partager, mais ce n'est pas la bonne méthode, c'est pas les bons moyens, mais sur le fond, nous arrivons, je crois à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire donner à chacun et à chacune sa place dans la société au travers du travail. Merci monsieur le ministre, la discussion générale est Close, la commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale de l'article 1er je suis saisi d'un amendement de monsieur le président, Canet. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est vrai que notre article 1er initiale pouvait non pas porter à confusion mais crée un émoi auprès des de ceux et celles qui soutiennent territoire zéro chômeur, nous nous sommes expliqués avec son président Laurent Grandguillaume avec les animateurs de cette association, je vous remercie Monsieur qui a pris toutes les dispositions pour avoir ces contacts utiles et la discussion, nous a permis de faire potentiellement évoluer cet article au au travers d'un amendement que j'ai l'honneur de vous présenter donc après cet échange avec le territoire zéro, chômeur de longue durée plutôt finalement que de généraliser cette expérimentation qui reste encore une expérimentation de manière anticipée à travers un dispositif que nous aurions voulu pérenne dans l'écriture initial de de notre texte, nous vous proposons donc de supprimer le plafond d'extension à 60 territoires et je puis vous confirmer qu'il y a plus de demandes que aujourd'hui ce nombre de 60 quand on recense exactement les initiatives au plan local, donc supprimé ce plafond de 60 territoires afin de permettre à tous les projets partenariaux territoriaux existant de venir intégrer cette expérimentation dans la mesure bien sûr, encore une fois, ou de répondre au cahier des charges, il est également proposé dans cet dans cet amendement de simplifier l'habilitation des nouveaux territoires par la prise d'un simple arrêté ministériel et non pas d'un décret comme le demande d'ailleurs l'association depuis longtemps, voilà donc l'esprit et le texte de cet amendement, madame la présidente. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, avec votre masque sur le nez. S'il vous plaît madame la la présidente, merci donc effectivement des territoires zéro, chômeur de longue durée, apparaît aujourd'hui comme étant le projet le plus innovants et prometteurs en matière de lutte conte le chômage de longue durée, prenant acte de cette expérimentation, l'article 1er vise à la transformer en un dispositif pérenne et accélérer son extension, les acteurs de l'expérimentation avec qui j'ai eu des échanges approfondis estime cependant qu'une généralisation est prématuré pour respecter le caractère de projet expérimental et la démarche du territoire au coeur des territoires zéro, chômeur de longue durée, cet amendement vise donc à remplacer le dispositif de l'article 1er par une suppression de la limite actuelle de 60, territoire, je rappelle qu'un décret en Conseil d'État est actuellement nécessaires pour y déroger dans le cadre de la 2ème phase d'expérimentation, outre la 19 territoires qui sont désormais habilités, le Fonds d'expérimentation qu'on veut le chômage de longue durée, recense 152 projets émergents en France, ainsi, tous ceux qui remplissent les conditions du cahier des charges pour être admis sans plus, attendent dans l'expérimentation par arrêté du ministre chargé de l'emploi, l'association Territoires zéro chômeur donc duré, qui considère que le nombre de sous son territoire doit être un minimum, soutient cette rédaction. L'avis de la commission est cependant défavorable. Merci, merci, monsieur le rapporteur, l'avis du Gouvernement, monsieur le ministre.

pour cette expérimentation sur 60 territoires d'ailleurs, c'était l'objet d'ailleurs de la réponse de la ministre Élisabeth Borne et de Brigitte Klinkert sur sur les 60, je crois que d'ailleurs ce que disait madame la sénatrice Frédérique Puissat il reste encore un certain nombre de choses à démontrer en la matière, ce n'est pas faire injure à l'expérience innovante, vous avez raison, monsieur le rapporteur, quel territoire ce jour que de leur demander aussi de poser les résultats et c'est pour ça que un comité scientifique qui a été mise en Oeuvres de manière à ce que nous puissions ont validé l'ensemble de ces résultats, on est dans cette démarche est une démarche de confiance vis-à-vis de territoires zéro chômeur et qui vient d'être construite et qui a été posée par une loi qui est toute récente, et moi je propose d'y rester, c'est pour ça que j'aurais un avis défavorable je le président. Merci, alors je vais mettre même pensé. Merci madame la présidente, le groupe écologiste soutient cet amendement car si l'assurance a été donnée par la ministre en CMP que le seuil de 60 expérimentation ne devait pas être compris comme un plafond, mais comme un plancher pouvant donner lieu à dérogation autant affirmer cela sans ambiguïté de façon non-discrétionnaire en supprimant ce seuil plafond au plancher, nous souhaitons établir que toute expérimentation sur un territoire qui seraient mature et respecterait le cahier des charges doit pouvoir candidater à l'habilitation, ce qui permettra d'ailleurs de mailler plus finement le territoire dans tous les départements, il pourrait y avoir des des expérimentations se confirme effectivement que, a priori, on parlait de 80, territoire expérimentation qui était mature et ça permettrait d'ailleurs d'enrichir l'évaluation dont vous parlez par la diversité des projets défendus. Merci, alors je vais mettre aux voix donc cet amendement j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission, je vous rappelle, s'il vous plaît, je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Alors voici le résultat du. Frutos numéro 109 sur l'amendement numéro 1 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 329 pour l'adoption 91 contre 238, le Sénat n'a pas adopté. je vais mettre aux voix l'article 1er, lequel je suis également. Saisi d'une demande de scrutin public par la Commission, il va donc être procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. D'accord, je suis même vote même vote merci beaucoup monsieur le président,

L'article 3 prévoit que les aides au titre d'un contrat aidé. Excusez-moi, dans le secteur non marchand ne peuvent être accordées que si le contrat porte sur des activités ayant pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion de ressources, il nous est apparu que limiter les CUI, CAE aux seules activités ayant pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion de ressources pourrait s'avérer trop restrictif et mettre en péril le fonctionnement de certaines associations qui accomplissent des actions utiles au lien social et qui répondent tout tout temps aux objectifs de la proposition de loi et donc afin de conserver ce levier volontarisme volontariste vers la conversion écologique des emplois tout en prenant mieux en compte les contraintes du terrain, nous proposons de remplacer cette conditionnalité par la possibilité de réduire l'aide au poste si les activités faisant l'objet du contrat n'ont pas pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion de ressources. Merci beaucoup, cher chers collègue l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci les madame la présidente, la conditionnalité environnementale introduite par cet article procède d'une démarche volontariste que je soutiens mes auditions cependant fait apparaître qu'elle pourrait être un facteur limitant, comme je l'avais proposé en commission cet amendement vise donc à remplacer cette conditionnalité par la possibilité de réduire l'aide au poste ses activités faisant l'objet du contrat aidé non pas leur non pas pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion de ressources, il me semble que cette solution est équilibrée et permet de remplir les objectifs de la proposition de loi sans compromettre le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire, cependant l'avis de la commission est défavorable à cet amendement. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, merci, on a le président, j'ai, j'ai un avis défavorable je m'en explique monsieur le Président, j'entendais monsieur le rapporteur, qui nous disait qu'il lui semblait que ça ça mettrait pas en difficulté, les autres pans de l'économie sociale et solidaire ou de l'insertion, je pense que ça va la mettre en difficulté, aujourd'hui on a près de 100000 contrats aidés qui sont signés par l'ensemble des collectivités, des associations sur d'autres périmètre que celui de la transition écologique, alors bien sûr on est favorable à ce que on puisse, dans notre pays, accompagner cette transition écologique mais je l'éditeur dans mon propos liminaire et je serai court Madame le président, parce que sur le fond, on a pris les moyens dans la loi climat résilience

Merci madame la présidente, nous le groupe écologiste va soutenir cet amendement, les écologistes ont toujours été attachés à la conditionnalité environnementale et sociale des aides publiques, rien d'anormal à ce que les aide à l'insertion professionnelle, accompagnent la transition écologique, compte tenu des besoins énormes et urgents sur chaque territoire cette relation d'ailleurs congruente se vérifie massivement 45 % des activités de l'expérimentation, 0 chômeur concerne la transition énergétique et écologique, la chercheuse Vabre dont j'ai parlé dans ma dit dans ma déclaration générale inclus, effectivement, la garantie d'emploi dans un plan national du prendre soin tant de la priorité du prendre soin de l'environnement que des individus en fait la dynamique partant des territoires s'oriente par elle-même, vers des activités sociales et soucieuse de l'environnement, ah si la Darès dans son étude de 2021 sur les expérimentations souligne que les entreprises à but d'emploi durant la crise sanitaire, par exemple, poursuit automatiquement se mobiliser pour s'investir dans des activités socialement utiles à leur territoire, que ce soit en matière d'équipement dispositifs sanitaires de base ou en terme de prise en charge des personnes les plus fragiles, donc la puissance publique reste légitime à aborder les employes participant cette ne s'est certes transition ou de façon peut-être plus positif d'acter que l'aide serait moins dans le sang des autres activités. Merci, cher collègue, alors je me mettre aux voix, donc l'amendement numéro 2 pour lequel j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Voici le résultat du scrutin numéro 110 sur l'amendement numéro 2 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 342 pour l'adoption 78 contre 264 le Sénat n'a pas s'adapter alors je vais mettre aux voix l'article 3 est ce que je peux considérer que c'est le même vote oui pour tout le monde, président Kanner oui donc même vote donc pas adoptée à l'article 4 l'amendement numéro 3. Même pour Merci madame la la présidente l'article 4 prévoit que les aides au titre d'un contrat aidé dans le secteur marchand ne pourront être accordées que si l'employeur a atteint la neutralité carbone ou s'est engagé, du moins dans la décarbonation ses activités, la proposition de faire du CICE, le vie des incitations à la décarbonation des modes de production et pertinente, afin d'accompagner la transition écologique tout en créant de nouvelles opportunités d'emplois mais pour ces contrats initiative-emploi nous souhaitons réservé cette conditionnalité de neutralité carbone aux entreprises de moins de 250 salariés parce qu'effectivement en dessous de ce seuil, les PME ne sont pas forcément capacité de produire des informations sur leur empreinte carbone, tels que le sens de notre amendement. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui merci madame la présidente, les contrats aidés dans le secteur marchand, peuvent être à la fois levier de créations d'emplois et d'incitation à la décarbonation des modes de production, l'article 4 va dans le bon sens en réorientant le contrat initiative emploi dans une perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre, toutefois il ne s'agit pas d'interdire de fait aux petites et moyennes entreprises de et de recourir aux contrats initiative emploi en faisant peser sur elle des coûts et une contrainte administrative prohibitifs, je rappelle que seules les entreprises de plus de 500 salariés où 250 salariés dans les Outre-Mer sont actuellement assujettis à l'obligation de réalisation d'un bilan carbone réglementaire cet amendement propose donc d'exonérer les entreprises de moins de 250 salariés de la condition de neutralité carbone prévue par l'article 4 cependant l'avis de la commission est un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre.

vous posant sur le sujet de la taille de l'entreprise, effectivement, disons, sur le fond, cette obligation de décarbonation je, je vais la faire peser sur les entreprises de plus de 150 salariés, je regarde le sujet des chiffres en fait acquis, à qui s'adresse ce type de contrat, essentiellement d'ailleurs aux TPE-PME, celles qui bénéficient de ces contrats, donc c'est vrai que. Lorsqu'on regarde le sujet des plus de 150 c'est presque un peu marginal en regardant c'est presque contre- intuitif, par rapport à votre objectif initial puisque vous allez perdre l'effet volume que vous cherchiez, au final, mais je ne vous reprocherai pas, sans doute, dans une volonté de rechercher un peu de consensus autour de cette proposition, je, j'avais envie de vous proposer d'autre chose, Monsieur le Président, canard c'est c'est de faire un peu de pub pour les dispositifs qui peut-être ne sont pas assez connu, la responsabilité en revient certainement au gouvernement, mais sur le fond, le volontariat territoriale en entreprise vers le VTT vers qui permet à des Pays-Bas ou des ETI de recruter des jeunes diplômés ou des étudiants pour les aider à se développer et à engager à s'engager sur la transition écologique, c'est aussi une forme de réponse et on a déjà dans leur arsenal sur le fond des réponses techniques qui permettent de d'aller dans le sens que vous souhaitez, je voulais aussi donner là un peu de perspectives à ma réponse défavorable sur votre amendement, on va dire qu'on peut partager aussi ses objectifs avec d'autres outils. Merci, Monsieur le Ministre, je vais mettre aux voix, donc l'amendement numéro 3 qu'a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté je mets vois l'article 4 pour lequel j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission fait procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos.

voici le scrutin, le résultat du scrutin numéro 100 sur l'article numéro 4, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs Hugot politique et notifié à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 329 pour l'adoption 76 contre 253, le Sénat n'a pas adopté alors à l'article 5 je suis aussi saisi d'un scrutin public, est ce que je peux considérer que c'est le même vote

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos.

le scrutin, le résultat du scrutin numéro 100 sur l'article numéro 4, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs Hugot politique et notifié à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 329 pour l'adoption 76 contre 253, le Sénat n'a pas adopté alors je suis saisi aussi d'un scrutin public pour l'article, c'est ce que c'est le même vote oui donc c'est le même vote donc pas s'adapter alors, mes chers collègues, je vais mettre aux voix l'article 7 si cet article n'était pas adopté, je considère très que le vote est le même pour l'article 8 il n'y aurait alors plus lieu de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur ces articles et sur l'ensemble, dans ces conditions, est ce que quelqu'un demande la parole pour expliquer son vote sur l'article 7 ans président canin. Madame la présidente merci, effectivement, vous avez bien fait de nous alerter, parce que sauf miracle dans cet hémicycle, mais je ne crois plus bien longtemps au miracle, nous allions tout droit vers la disparition totale de cette proposition de loi, ce que je regrette bien évidemment quelques mots globalement dire à nos collègues de de la droite de l'hémicycle que ben, on est content de vous retrouver bien la droite sur vos positions, j'ai entendu parler de socialisme fiscal mais il est vrai que ça fait bientôt 10 ans que vous n'êtes plus au pouvoir je crains d'ailleurs que Douglas me l'a dit tout à l'heure, ça risque de continuer donc dans ce cadre, soyez innovants, je vous le dis avec beaucoup de de dire la d'amitié presque soyons, soyons innovants comme nous pouvons l'être en la matière, monsieur le ministre, et aussi pour bien sûr pour la majorité de la commission, qu'est ce que nous voulions faire ce soir avec un succès d'estime bien évidemment que nous prévoyons, nous voulons donner un message finalement à celles et ceux qui aujourd'hui sont plus qu'au bord du chemin, ils sont même dans dans le fossé et depuis de nombreuses années de génération en génération population qui aujourd'hui ne demandent qu'à être reconnu, ce qui ne sera pas le cas ce soir. Vous avez toujours porté, monsieur le ministre vous et et et ce qui vous entoure l'idée du ruissellement du 1er de cordée l'idée que la main invisible du du du marché les pouvoir tout réguler et vous avez découvert que finalement il y avait des fractures dans notre pays, celles des gilets jaunes, celle de laissés-pour-compte de la crise sanitaire et qu'il fallait leur répondent avez même découvert parfois des mesures quasiment keynésienne, mais le dos dans les cordes, parce que vous ne pouviez pas faire autrement, nous, ce n'est pas notre conception nous croyons à la force de l'État et nous croyons à l'intervention de l'État pour tendre la main à celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin de solidarité, c'était le sens de cette PPL qui va prospérer sur d'autres milieux plus politiques dans le cas de cette élection présidentielle, je regrette que aucun de nos arguments n'est peut-être qu'on n'ait pu être pardon prise en considération ce soir mais nous continuerons notre combat. Merci. Merci. Je vais donc mettre aux voix. L'article 7 pour lequel j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission, il va être donc procès de scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

ouvert. Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos.

Donc un petit problème, donc je vais vous donner les résultats du du scrutin, nombre de votants 343 exprimés 329 pour 91 contre 238, le Sénat n'a pas adopté l'article 7 et donc rejetée, il en est donc de même de l'article 8 un vote sur l'ensemble n'est donc pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte en conséquence, la proposition de loi n'est pas adopté. madame la présidente. par rapport au président Kanner salue néanmoins le travail des rapporteurs, c'était simplement pour dire : Monsieur le Ministre, puisque c'est notre dernière séance vous remercier du travail que nous avons accompli ensemble, nous n'avons pas été toujours d'accord sur des textes, mais je voulais saluer néanmoins ce travail et remercie également votre cabinet pour ces mois de travail en commun. Merci beaucoup monsieur le rapporteur. merci madame la présidente, je voulais aussi à mon tour remercier des administrateurs qui m'ont accompagné tout au long de ces auditions et puis remercier, madame la présidente de la commission et des membres de la commission, M. vous me, je ne le le ministre pour Merci. Monsieur le ministre, je voudrais courbe la main le président juste à la fois remercier, madame la présidente, monsieur le rapporteur pour leurs propos à mon égard et aussi à l'égard de mon cabinet, dire : Madame le président, que c'est toujours un plaisir de venir travailler au Sénat avec l'ensemble des sénatrices et les sénateurs pour à la fois la la qualité des débats, on peut effectivement exprimer des avis opposés parfois les uns aux autres, mais le faire avec une tranquillité d'esprit, qui d'ailleurs, je crois, enfin ce qu'il se débat démocratique dire au président que je je crois moi à la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, je crois que les 2 sont utiles dans la vie et je pense que les solutions parce que sur le fond, je crois que nous nous avons les mêmes objectifs en la matière, c'est de ne laisser personne au bord du chemin dit dans le fossé, c'est bien ce que j'ai essayé moi ne vous partagez pendant 7 heures et demie de débat merci madame le président. Merci monsieur le ministre, je ne vais pas suspendre la séance ça et demandé à chacun de laisser les places qui sont ici pour que ministre suivant puisse arriver mais Staquet et puis que chacun puisse pas sa place aussi au niveau de la Commission, merci.

l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à maintenir le versement de l'allocation de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses du parent bénéficiaire, présenté par Madame Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues dans la discussion générale, la parole est à madame la présidente, Laurence Rossignol, auteur de la proposition de loi et pour 10 minutes. Plaît, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure chers. Collègues écoutez, je suis très heureuse de vous proposer cette proposition de loi dernière proposition de loi de cette législature, elle se situe entre la Saint-Valentin et le 8 mars il n'y avait pas meilleure date pour une proposition de loi visant à maintenir le versement de location de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses, cette proposition de loi que ma collègue Michèle Meunier va rapporter dans quelques instants et courte 2 articles et les simples, elle vise à supprimer un alinéa de l'article 523 2 du code de la Sécurité sociale, elle est surtout à mes yeux un volet de ce que devrait constituer une politique globale de soutien aux familles monoparentales et qui inclurait la fin de l'imposition des pensions alimentaires le prolongement jusqu'à 12 ans d'un complément mode de garde spécifique et la mise en place d'un délai avant le retrait des majorations des prestations sociales soumise à conditions d'isolement notre politique familiale dont nous pouvons être fiers et caractérisé, entre autres, par sa grande souplesse d'adaptation aux évolutions de la société, elle accompagne par exemple rail des femmes par le soutien aux modes d'accueil à l'accueil des jeunes enfants, crèches, assistantes maternelles et là progressivement substituer la notion de parents et de parentalité à celle de famille elle est neutre à l'égard des formes de familles car elle est centrée sur l'enfant et sa protection. Près d'un quart des familles sont désormais composé d'un seul parent et dans 80 % 82 % des cas ses parents se parent est une femme, c'est la raison pour laquelle je parle souvent de mère monoparentale, bien entendu, toutes ces mères monoparentales ne sont pas en situation d'isolement, d'absence de pension alimentaire beaucoup reçoivent une pension alimentaire, fort heureusement, ou encore de pauvreté, mais néanmoins sur les 4 millions d'enfants qui vivent dans une famille monoparentale 1,4 1000000 d'entre eux vit en dessous du seuil de pauvreté, il y a donc une nécessité à aider les familles monoparentales pour protéger les enfants et les protéger, surtout de la pauvreté. J'évoquais il y a un instant l'agilité et l'adaptabilité de la politique familiale. Je prends comme exemple la transformation en 1984 de l'allocation orphelin en allocation de soutien familial, cependant, la suspension du versement de cette allocation en cas de remise en couple, que le couple soit formel ou informel. Du parent bénéficiaire me paraît aujourd'hui anachronique et dans l'esprit que j'évoquais il y a une seconde d'adaptabilité constante de la politique et des prestations familiales à l'évolution de la société, il me paraît maintenant le moment venu, de supprimer cette suspension de l'allocation de soutien familial lorsque le parent bénéficiaire a un nouveau couple construit un nouveau couples. En fait, cette suspension de l'ASF en cas de remise en couple et je précise bien que le couple peut être formel ou informel, part d'un postulat ce postulat, c'est celui de la création d'une nouvelle solidarité infra-familiales avec un nouveau conjoint grâce au nouveau conjoint par le nouveau conjoint, alors que, et je vais citer la le rapport conjoint de l'Inspection générale des finances. Et de l'Inspection générale des affaires sociales, qui a été remis en juillet 2021, ce rapport dit que cette solidarité intrafamiliale lié à une nouvelle remise en couple est loin d'être systématique, il est en effet fréquent que le nouveau compagnon soit lui-même séparé et quitte une pension alimentaire qu'il verse à la mère de ses enfants quand elle en a là qui en Et par ailleurs je souhaiterais attirer votre attention sur une incohérence qui me paraît importante. Lorsque un parent séparé. Je perçois une pension alimentaire du père de ses enfants, de son ex-conjoint cette pension alimentaire et versez-y compris. Kant se parent se remet en couple, le juge aux affaires familiales ne va pas décider que le blé, la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants qui est acquitté par le parent séparé est prévu par la convention. Est suspendue ou retirée au motif que la mer à un nouveau conjoint, on continue de verser la pension alimentaire, lorsque la mer se a un nouveau couple se crée une nouvelle famille. Mais lorsque. Il n'y a pas de pension alimentaire parce que le père est défaillant parce que il est insolvable, parce qu'il n'existe pas, parce qu'il a disparu dans les cas verse dans la le profil des bénéficiaires de l'ASS, il y a les enfants orphelins, il y a les enfants nés sans filiation paternelle identifiée et puis a les enfants ayant une filiation mais dont les pères n'assume pas la pension alimentaire, donc c'est la solidarité par la Caisse d'allocations familiales qui vient se substituer aux pères défaillants et dans ce cas-là, on suspend le versement de l'allocation, il y a là une incohérence sur lequel j'attire votre attention et il est bien entendu qu'il ne viendrait à l'idée de personne de proposer que on ne verse plus la pension alimentaire encadre remise en cours. Le maintien de l'ASF après. Remise en coupe n'est pas une idée totalement nouvelle, c'est une idée qui avait déjà été expérimentée en 2014, alors je prends une toute petite parenthèse historique parce que comme monsieur le ministre, qui lui aussi est très content de nous voir pour la dernière fois dans cette législature.

pour nous faire tout le bilan de toute la politique du gouvernement au cours des 5 dernières années, et d'ailleurs, tout est prêt et qu'il va nous expliquer tout ce que le gouvernement a fait pour les familles monoparentales, avant même qu'il le fasse un petit rappel historique. La garantie des impayés de pensions alimentaires a été créé, expérimenté en 2014, parce que tout n'a pas commencé en 2017 comme j'entends parfois dans bien des domaines elle a été créée, expérimentée en 2014 généralisé en 2016 et l'Aripa, l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires a été créé en 2000 17 mai début 2017 en janvier. Et après, le gouvernement et je l'en remercie, a poursuivi sur cette lancée et en et approfondie, ce qui avait déjà été posée et les fondations étaient là pour faire encore plus et mieux, et quand tu nous avons fait en 2014 la garantie un bide, pension alimentaire, nous avions prévu le maintien pendant 6 mois du versement de cette Qui êtes sous forme expérimentale et au moment de la généralisation la techno-structure c'est mobiliser fortement pour faire supprimer.

n'a été donnée à s'inspirer de cette expérimentation, nous n'avons jamais pu savoir par la technostructure, si elle avait été conclu en tout pas concluante mon point de vue, c'est qu'elle était concluante, mais vous savez, il y a parfois une force technocratique qui s'impose à tous, a été le cas, donc je vous raconte ça pour vous dire que c'est pas une idée totalement farfelue qu'elle a déjà expérimenté, et que les éléments qu'on a pu avoir dans les CAF étaient positif, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reviens vers vous avec mes collègues pour vous demander de continuer de faire évoluer notre politique familiale alors je sais que les collègues de la droite aimerait une grande réforme de la politique familiale, je ne crois pas aux grandes réformes de la politique familiale, ça ne s'est jamais produit comme ça. Pour différentes raisons, la politique familiale, elle évolue avec la société, elle s'adapte en permanence et je ne suis pas sûr de souhaiter une grande réforme de la politique familiale, par ailleurs, tellement je ne suis pas certaine non plus que les fondamentaux. Que nous partageons sans doute en nombre serait respectée dans cette grande réforme libérale des politiques familiales qui pourrait tout à fait voir le jour dans le l'ambiance dans l'air du temps, dans lequel nous sommes aujourd'hui alors, à défaut d'une grande réforme, je vous propose mes chers collègues, d'adopter une petite réforme essentielle pour les familles monoparentales, une réforme qui met fin à un anachronisme et une effort réforme qui peut également poser les fondements d'un grand plan en faveur des familles monoparentales, je vous remercie.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le groupe socialiste, écologiste et républicain, a demandé l'inscription à l'ordre du jour dans son espace réservé de la proposition de loi déposée par notre collègue Laurence Rossignol, visant à maintenir le versement de l'allocation de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses du parent bénéficiaire, je ne m'attarderai pas très longtemps sur l'article 2 de ce texte, il s'agit en effet d'une demande de rapport au gouvernement sur la diversité des situations familiales et leur prise en compte sur notre régime fiscal, un quart des familles françaises, on le sait, sont désormais monoparentale, contre 12 % en 1990 plus largement les modèles familiaux qui ne saurait dorénavant se résumer à la famille nucléaire ou les façons de faire famille évoluent, si bien qu'engager une réflexion sur l'adaptation de notre fiscalité à ces changements me paraît essentiel. C'est pourquoi je suis personnellement favorable à l'adoption de cet article, toutefois, fidèle à sa position sur les demandes de rapport, la commission de notre Sénat a rejeté cet article, j'en viens donc à l'article 1 en revanche qui lui porte sur le dispositif ambitieux promu par ce texte, il propose de ne plus conditionner le versement de l'allocation de soutien familial à l'isolement du parent bénéficiaire l'allocation de soutien familial est une prestation de la branche famille versées sans condition de ressources à un public spécifique, elle est accordée à plus de 800000 foyers en 2021 pour l'éducation des enfants, privé du soutien d'au moins d'un parent 7 1 1000000 300 1000 enfants qui en sont bénéficiaires, son montant forfaitaire pour chaque enfant, 116 euros est accordé si l'enfant est privé de l'aide d'un de ses parents et 155 euros, si les 2 parents sont absents, l'allocation de soutien familial a pris le relais en 1984 de l'allocation orphelin et englobe désormais des situations beaucoup plus diverses que les seuls enfants de parents décédés, elle est versée à la personne ayant la charge d'un enfant dont la filiation n'est pas établie au regard d'au moins un des parents, elle permet également de remplacer la pension alimentaire, si un des parents de l'averse pas où est reconnu comme hors d'état de de faire face à son obligation en raison principalement de son insolvabilité, dans le cas où le parent se soustrait même partiellement à son obligation de versement de la créance alimentaire l'ASF est versée à titre d'avance aux parents créanciers, à charge pour la Caisse d'allocations familiales de recouvrer la pension alimentaire auprès du parent débiteur un vaste mouvement de réformes engagé depuis 2014 ça a été rappelé, et merci Laurence Rossignol d'une mettre les pendules à l'heure en 2014 donc contre les impayés de pensions alimentaires, ce qui a permis de monter en charge de cette allocation sociale familiale recouvrables enfin depuis 2016, l'ASF différentiel permet de compléter la pension alimentaire, si cette dernière est fixée à un montant inférieur à celui de l'ASF en parallèle à ces critères d'éligibilité, le parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant reçoit l'allocation de soutien familial, sous strictes conditions d'isolement, l'allocation cible donc les seules familles monoparentales et cesse d'être versés si l'Europe le parent reprend une vie commune, quel que soit son statut Mariage, Pacs, concubinage, selon la Caisse nationale des allocations familiales, environ 24600 par an auraient ainsi perdu le bénéfice de l'ASF non recouvrables en 2020, parce qu'ils ont choisi de se remettre en couple, de prime abord ce ciblage pourrait paraître fondée en raison de la surexposition des familles monoparentales, à la précarité, je vous rappelle que 40 % des enfants vivant dans une famille monoparentale sont considérés comme pauvres, selon l'Insee, les dépenses d'ASF, qui s'élevait à 1 milliard 79 millions d'euros en 2020 sont donc essentielles pour ces familles, néanmoins, en faisant perdre le bénéfice de l'ASF aux parents qui se remettent en couple, la condition d'isolement l'emporte de nombreux effets pervers : elle est source d'incohérences et par conséquent d'incompréhension pour les familles concernées, tout d'abord cette condition dissuade certains parents isolés de reprendre une vie commune avec un conjoint par crainte de remettre en cause l'équilibre fragile de leurs finances 70 % des bénéficiaires de l'ASF appartiennent aux 2 premiers déciles de la redistribution des revenus, les familles monoparentales, aux revenus les plus modestes sont même plus nombreuses à recevoir une ASF qu'une pension alimentaire et la perte de 116 euros par enfant n'est donc pas négligeable pour ces familles précaires dont une partie, choisi de sacrifier ses projets de vie conjugale ou marital pour des raisons matérielles. Du point de vue de l'efficacité des politiques publiques ce découragement à sortir de la monoparentalité est d'autant plus regrettable qu'en moyenne le niveau de vie des parents isolés augmente après la remise en couple, en reprenant une vie commune, ces personnes peuvent réaliser des économies d'échelle sur les charges de la vie courante, elles peuvent également concilier leur vie familiale et professionnelle en abandonna en abandonnant certains fardeaux de la monoparentalité aussi la remise en couple peut-elle favoriser la reprise d'une activité professionnelle, alors que 35 % des parents isolés sont sans emploi, agit ainsi comme une barrière maintenant maintenant les familles dans une trappe à isolement et plus encore une trappe à pauvreté, s'agissant des familles ayant tout de même choisi de se remettre en couple, la perte de l'allocation de soutien familial réduit mécaniquement leur autonomie financière au sein de leur nouveau ménage les parents isolés, dont je répète 82 E % sont des mères risquent de se retrouver dans une relation de dépendance à l'égard de leur nouveau conjoint pour l'éducation et l'entretien de leurs propres enfants, cette situation n'est pas souhaitable en soi, de plus, ce serait un postulat erroné que de considérer que le nouveau conjoint contribuent systématiquement aux frais de l'entretien de l'enfant, il n'y ait tenu par aucune obligation juridique, surtout en dehors, en par ailleurs il peut lui-même avoir des enfants à charge et disposer de revenus modestes, voire être aussi un ancien parents isolés ayant perdu le bénéfice de l'ASF, enfin la restriction du bénéfice de la assaut de l'allocation de soutien familial au seul parent isolé ne se justifie pas du point de vue de l'intérêt supérieur des des enfants quel que soit le statut marital ou conjugal du parent avec lequel ils vivent, il demeure privé du soutien du second par an, la condition d'isolement s'appliquant au versement de l'allocation n'a donc aucune raison d'être, la perte de l'ASF au bénéfice de leur éducation et d'autant plus incohérente que les parents créanciers qui se remettent en couple ne voit pas pour autant leur droit à une pension alimentaire être suspendu cette différence de traitement pénalise les bénéficiaires de l'ASF, alors même qu'il se trouve dans une situation de plus grande vulnérabilité pour toutes ces raisons, la suppression de la condition d'isolement apparaît comme nécessaire, elle a d'ailleurs été recommandée par le Haut Conseil de la famille de l'enfance et de l'âge, dans son rapport du 28 septembre dernier bien entendu d'autres paramètres des dispositifs en faveur des familles ou nos parental mériteraient d'être réformés dans une approche plus globale, je pense notamment à la prise en compte inégal des pensions alimentaires et de l'ASF dans les bases ressources des prestations sociales ou de l'impôt sur le revenu, ce traitement différencié rend paradoxalement préférable le versement d'une ASF plutôt qu'une pension alimentaire, il n'en demeure pas moins qu'en maintenant le versement de l'allocation aux parents éligibles qui ne remplissent plus la condition d'isolement, nous avons la possibilité d'adopter la une mesure de bon sens, sans attendre une réforme d'ampleur de la politique familiale dans sa globalité, vous aurez donc compris mes chers collègues, qu'à titre personnel, je suis favorable à l'adoption de l'article 1er de cette proposition de loi, la commission des affaires sociales n'a toutefois toutefois pas adopté cet article, ni même la proposition de loi et c'est donc le texte initialement déposé par l'auteur que nous affréterons à examiner tout à l'heure je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Adrien taquet secrétaire des. Sa chargée de l'enfance et des familles.

Madame la présidente, madame. La présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure. Madame la sénatrice Rossignol mesdames et sénatrices, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis ce soir. Avec plaisir. De vous voir. Tout court. Comme ça a été le cas depuis le le début de cette mandature pour examiner cette proposition de loi qui vise à maintenir le versement de l'allocation de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses du parent bénéficiaire allocations dont vous contestez madame la rapporteure, le mécanisme de suspension puisqu'il imposerait au parent bénéficiaire et je je cite l'exposé des motifs de choisir entre la solitude et la dépendance économique alors avant même de revenir sur le fond de votre proposition, je tiens à rappeler. Le gouvernement partage pleinement votre occupation de soutenir les parents isolés en répondant au mieux et durablement à leurs besoins et j'aurai l'occasion oui Madame Rossignol, vous l'avez évoqué d'y revenir plus tard, en détaillant les mesures spécifiques déployés par ce gouvernement depuis maintenant 5 ans, et vous verrez que j'adresserai également quelques perspectives pour l'avenir en cette période particulière. C'est bien sûr indispensable quand on sait que les familles monoparentales qui représente, aujourd'hui, vous l'avez dit, l'une et l'autre, plus d'un quart des foyers sont pour plus d'un tiers d'entre elles, en situation de précarité en ce qui concerne tout d'abord votre idée de maintenir le versement de l'allocation de soutien familial pour le parent bénéficiaire en cas de remise en coupe par Pacs, mariage, concubinage je considère Madame la rapporteure qu'elle aurait pour première fait de vider cette prestation de son sens je crois. Et pour second effet de brouiller l'ensemble de notre politique familiale, l'ASF a été créé, vous l'avez rappelé en 1970 en remplacement de l'allocation aux orphelins dans le but de soutenir les personnes qui assument seules la charge effective et permanente d'un enfant de moins de 20 ans privés de l'aide, l'un de ses 2 parents. Une allocation créée pour aider financièrement les parents isolés changeraient donc de nature avec votre proposition dans un sens qui me semble à la fois peu justifier socialement risquée juridiquement. Peu cohérent avec notre système de prestations familiales et enfants financièrement coûteux peu justifier socialement tout d'abord, car la remise en couple restaure les économies d'échelle qui avait disparu à la suite de la séparation, ce sont les données de l'Insee qui le démontre, le taux de pauvreté des enfants et de 40,5 % pour ceux qui vivent avec un seul parent lorsqu'il n'est que de 15 que de 15,5 % pour les enfants dont les parents sont en couple. Juridiquement risqué ensuite. C'est ce qu'elle conduirait les couples dont l'un des membres a été préalablement situation monoparentale a bénéficié d'un montant de prestation supérieurs aux couples non préalablement séparés. Différence de traitement entre les couples qui me paraît difficilement défendable et qui serait probablement constitutif d'une rupture d'égalité risqué, je dirais, juridiquement, donc, mais aussi budgétairement, il faut rappeler que l'ASF n'est pas une prestation sous conditions de ressources. La suppression de la condition d'isolement entraînerait une hausse significative du nombre des bénéficiaires de l'allocation pesant nécessairement la question du coût d'une telle réforme, et donc de son financement, on vient de rayon nous à faire le choix de subordonner le bénéfice de la prestation est une condition de ressources qui n'existe pas aujourd'hui, je ne pense pas cela souhaitable. Ces 2 risques à la fois juridique et budgétaire sont du reste d'autant plus grand que si nous suivions la logique qui est la vôtre, il s'en suivrait rapidement que tous les autres dispositifs favorables aux familles monoparentales devraient eux aussi être étendu au-delà de la remise en cours. Je pense ici la majoration du montant et du plafond du complément de mode de garde, la majoration du plafond de l'allocation de base et des primes à la naissance et à l'adoption de la page ou encore à la majoration du plafond du plafond du du complément familial. Il me semble enfin également qu'une telle évolution brouillerait je l'évoquais la lisibilité de notre système d'aide quelle différence ferait-t-on en effet entre une ASF versées à des familles monoparentales ou en coupe et les prestations familiales qui ne nécessite pas de conditions d'isolement et vise à couvrir les dépenses d'entretien des enfants. Et en l'absence de grandes différences alors pourquoi 2. C'est C'est là, je pense que le risque le plus pernicieux, car vous voyez qu'en en tirant le fil votre proposition pourrait conduire certains à considérer que ces dispositifs spécifiques aux familles monoparentales mais qui serait étendue aux familles, ex-monoparentales remise en couple ne font que doublonner le droit commun à toutes les familles, il s'en faudrait alors de peu pour que les mêmes en appelle à leur suppression et je pense que nous serons d'accord pour considérer que cela n'est pas souhaitable évidemment ou encore au retour de la situation à la situation initiale dont le détour aura permis de constater qu'elle était, dès le début, équilibré, en conclusion, madame la rapporteure. L'article 1er de cette proposition de voix me semble proposer une solution inadaptée à un problème qui lui, pourtant, est bien réelle, à savoir celui de la fragilité des familles monoparentales. Nous sommes déjà beaucoup mobilisé pour elle, mais à chaque fois que nous pourrons encore amplifier notre action en leur faveur, nous le ferons. Tout d'abord, et pour conclure, s'agissant de l'ASF, le principal sujet et selon moi, celui de son taux trop élevé de non-recours. En effet, une étude menée par la cave de Gironde en 2018. à démontré qu'environ 15 % des bénéficiaires potentiels de l'ASF, ni recouraient pas, ce sont donc près de 200000 foyers qui seraient concernés au niveau national, c'est un taux de non recours très élevé qui doit nous préoccuper, nous conduire à mobiliser de nouveaux moyens pour détecter les bénéficiaires potentiels est allé à leur rencontre, cela passe notamment. Par le déploiement de des dispositifs dits de Data Mining, qui permettent, sur la base de recoupement de données de détecter les familles potentiellement concernés, la CNAF a déjà initié cette démarche sur la base de ses propres données, elle pourra prochainement le faire avec les informations d'autres organismes de Sécurité sociale un décret en ce sens devant paraître d'ici le mois de mai. De la même manière, les CAF et le MSA développe des parcours spécifiques pour les familles en fragilité, vous le savez, qui permettent de procéder à des détections de droit auxquels les foyers ne savent parfois même pas qu'ils peuvent, ils prétendent. Nul doute que le déploiement de ce type de service constituera un axe fort de la prochaine la prochaine cause entre la CNAM et l'État dans l'lait. Concertation négociations vont commencer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Au-delà de ces évolutions, il s'agira à l'avenir d'amplifier les actions en faveur des familles monoparentales, que nous avons mis en oeuvre dès le début du quinquennat Que des mesures avaient pu être prises avant même le début de ce quinquennat. Je pense tout d'abord pour vous rejoindre madame la sénatrice Rossignol au service public des pensions alimentaires dont vous avez rappelé la genèse. Que je connaissais en dépit de la jeunesse en politique. Qui permet aussi bien d'assurer le versement intermédiés des pensions que leur recouvrement en cas d'impayés en effet pour une femme par pour un homme aussi un défaut de paiement, ça n'est pas qu'un accident comptable, ce n'est pas qu'un sujet de trésorerie ce type d'insécurité financière peut-être un véritable drame qui plonge des familles des enfants dans la pauvreté, aujourd'hui, le service d'intermédiation fonctionne, plus de 60000 personnes ayant déposé une demande. Mais ces personnes ont, de leur immense majorité déjà vécu un impayés de pensions alors même que notre objectif est d'intervenir avant, avant tout pays, dans un objectif de prévention. Pour aller plus loin pour mieux protéger, nous avons décidé de généraliser cette intermédiation avec vous puisque vous l'avez fauté. Dans Dans le cadre de la de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, et dès le 1er mars dans quelques jours, elle sera systématiquement mis en place lors de la fixation de la pension par le juge, hormis lorsque les 2 parents le refuse expressément, c'est un système, vous le savez, vous le connaissez bien dont l'efficacité a été prouvée au Québec et je forme le voeu que la prochaine période. Dans laquelle nous sommes désormais nous donne l'occasion de poursuivre sur le chemin de l'adaptation de notre politique à cette réalité familiale qui est la gestion de l'après-séparation. Car plusieurs questions cruciales me semble rester posée en dépit des efforts considérables consentis et des progrès majeurs accomplis ces dernières années, il s'agira selon moi notamment, d'une part, de parfaire encore la garantie de recouvrement des pensions et de reconsidérer très probablement le niveau de notre soutien aux plus modestes d'entre elles. De mettre ensuite sérieusement à l'étude, la question de l'adéquation entre les règles de partage des aides familiales et les réalités vécues par les familles. Enfin, à cette occasion, probablement de mettre au clair ce qui resterait à l'être, s'agissant de l'étendue des devoirs de solidarité conjugale à l'égard des Besançon. Je pense aussi à nos aides à la garde d'enfants, des filles pour toutes les familles casse-tête trop souvent insoluble pour les familles monoparentales, en particulier. Nous avons pris des mesures fortes en la matière, avec en particulier, vous le savez la majoration de 30 % pour les familles monoparentales du montant du complément de mode de garde en 2018. Je rappelle également que 2 millions d'euros supplémentaires ont été votées par la CNAF au printemps 2021 pour soutenir financièrement des centres de loisirs sur des horaires élargis, de 18 heures pour faire en sorte que dans les territoires où les trajets domicile travail sont très longs, par exemple en seconde couronne. Les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes de la fin des cours jusqu'au retour de leurs parents à la maison. Ce sont ainsi 580000 nouvelles heures d'accueil en soirée qui seront financés à hauteur de 80 % jusqu'à la fin de cette année 2022. Et il nous faudra je pense demain aller plus loin et achevé la construction entamée d'une société plus accueillante pour les familles, pour toutes les familles. Car nous voulons garantir à toutes les familles, l'accès à des congés à des services à la fois mieux adapté à leurs aspirations, mais surtout essentiel pour la l'organisation de leur vie quotidienne. L'universalité des services aux familles, elle est attendue. Et peut-être, probablement, très probablement encore plus par les familles monoparentales que par les autres. Elle permettra non seulement de mieux les protéger de la pauvreté en complément des aides familiales mais aussi et surtout de leur donner les outils pour s'en prémunir durablement par elle-même, par exemple, ou en se formant, en prenant, ou en reprenant un emploi, c'est l'horizon que le président de la République a tracé et auquel le Conseil économique, social et environnemental travaille à ma demande d'un droit garanti un accueil du jeune enfant à un prix raisonnable et similaire par une assistante maternelle ou en crèche. Ou que l'on se trouve sur notre territoire, c'est aux familles monoparentales avant tout que bénéficiera cette révolution. Car cela on sera une du droit à la garde d'enfants, dans notre pays, enfin consacré dames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis fier d'avoir donné aux familles monoparentales toute leur place dans notre politique familiale, dans la lignée totalement assumé de ce qui a pu faire auparavant, j'ai confiance que nous poursuivrons demain dans cette voie, madame la rapporteure, vous partagez cette ambition et j'en suis heureux nous divergeons sur votre proposition et j'en suis Marie. Mais ensemble sachant peut-être parfois nous garder de mesures trop vite. Imaginée et conçue et concentrons nous concentrons nos efforts sur les problèmes concrets des familles qui nous reste à résoudre, faciliter la la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle, ainsi que leur accès à l'emploi, concevoir des offres nouvelles qui puisse alléger leur charge mentale avec des solutions de répit, faire en sorte que toutes familles monoparentales puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie, pour cela, vous me trouverez toujours à vos côtés, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Alors, dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame la rapporteure générale Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre madame la rapporteure, chers collègues, en préambule, je voudrais simplement rappeler que le 1er objectif assigné à la politique familiale française et de compenser les charges de famille selon une logique de redistribution horizontale en réformant au coup par coup, année après année, rabotage après rabotage les aides aux familles ont perdu leur cohérence cette cohérence souffre d'un empilement d'aide disparates aux conditions d'attribution, variables, ces dispositifs sont donc devenues souvent illisibles pour le commun des mortels, ce qui tend à les rendre moins efficace, crée des inégalités de situation et parfois des phénomènes d'échappement et comme ça a été dit de non-recours. Lorsque j'étais rapporteur de la branche famille au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, j'ai à de multiples reprises regretté le manque d'ambition de notre politique familiale qui s'est contenté d'être la variable d'ajustement des politiques budgétaires des gouvernements successifs. Je remercie donc madame Laurence Rossignol, qui par le biais de sa proposition de loi permet de mettre à l'agenda, la situation des familles monoparentales qui représentent, comme ça a été dit par Madame la rapporteure 25 % des familles aujourd'hui et plus largement de débattre de notre politique familiale. Il est urgent de redonner un vrai souffle à la politique familiale au-delà du renforcement de quelques dispositifs ciblés, elle devrait évoluer qualitativement vers l'accompagnement de chaque enfant, soit dit en passant, l'ouverture du droit aux allocations familiales dès le 1er enfant me paraît être une piste à développer sérieusement et c'est ce qui a été proposé par mon collègue Olivier Henno. J'en reviens à la proposition de loi présentée ce jour. Beaucoup d'incompréhension et à raison perdure autour de l'attribution ou non de l'allocation de soutien familial, contrairement à la pension alimentaire, les droits à l'ASF sont interrompues lorsque le parent bénéficiaire fait état d'une nouvelle situation de vie conjugale ou marital cela génère donc un fort sentiment d'injustice et vous l'avez très bien exprimé cependant, il faut bien comprendre que la question de la pension alimentaire est un effet de la séparation du 1er couple et son versement doit être réglé avec le payeur, l'allocation de soutien familial venant simplement en garantie lorsque le payeur ne peut plus la payer cette forme d'ASF agissant telle une garantie à transformer la fonction initiale de l'ASF, qui visait les orphelins, cela a généré une confusion certaine. Il est utile de rappeler que les enfants mineurs vivant en famille monoparentale sont 2 fois plus touchés par la pauvreté, que l'ensemble des familles, soit plus de 40 % d'entre eux, et je pense que nous sommes tous effectivement très insatisfaits de cette situation. Ces chiffres démontrent ainsi tout l'enjeu économique que revêt la situation amoureuse du parent ayant la charge de l'enfant. Face à cette réalité : la perte de l'allocation de soutien familial peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis du nouveau partenaire. Aussi la proposition de loi qui nous est soumise et pertinente de ce point de vue. Je regrette que le texte aborde la question de l'ASF, s'en remettre à plat ce qui a été identifié comme étant problématiques pour la Cour des comptes. C'est-à-dire clarifier le dispositif en prévoyant des dispositions particulières pour les orphelins ou pour les enfants dans le lien de filiation n'est pas légalement établie avec le second par an et d'autres dispositions dans les autres cas. Une autre voie certainement coûteuse, aurait été de proposer dans le texte initial, une revalorisation de l'allocation qui est actuellement de 116 11 euros de l'enfant, voire de l'indexer sur un pourcentage du SMIC. En effet, lorsqu'il s'agit de remplacer une pension alimentaire peut-on aujourd'hui considérer que le montant de l'allocation est suffisant. Pour conclure, nous considérons qu'il existe bien un sujet à éclaircir et nous avons entendu les demandes des associations toutefois nous considérons au groupe Union centriste que cette proposition de loi en ouvrant pas l'ensemble du sujet, propose une solution incomplète. Nous aurions préféré étudier un texte réformant plus en profondeur le sujet voire posant la question de l'interaction. De l'ensemble des prestations afin d'envisager les aides sociales à la famille dans leur globalité, par conséquent, le groupe Union centriste s'abstiendra. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes. Madame la présidente, madame, monsieur le ministre madame la rapporteure, chers collègues, faut-il maintenir le versement de la location de ce de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses du parent bénéficiaire, voilà la question qui nous est posée, aujourd'hui, je tiens à remercier nos collègues du groupe socialiste pour cette proposition de loi qui nous permet de parler de ces familles monoparentales dont on ne parle que trop peu en effet à une situation familiale, souvent difficile s'ajoute une situation financière délicate avec à 82 % des cas une mère souvent contraintes à une activité partielle, donc précaire et des revenus faibles par ses conditions d'octroi, l'allocation de soutien familial est une aide conséquente et souvent primordial pour les plus de 800000 familles concernées. Le débat sur son individualisation mérite d'être soulevée par les difficultés que cette allocation peut poser sans réel, il y a d'abord la perte de revenus engendrée suite au retour d'une vie à un couple qui représente qui toucherait 24000 par an, je partage complètement les propos de la rapporteur lorsqu'elle indique que cela peut constituer un frein à une remise en couple, le manque à gagner parfois trop importante pour ces familles qui appartiennent dans la large majorité d'États ou d'ici là, les plus faibles, les situations dans ces situations, les nouveaux conjoints participent à la vie à l'éducation et à l'assistance financière de l'enfant le nom: maintien de l'ASF lors d'un retour à une vie de couple peut même aggraver la Vullnet la vulnérabilité de ces familles qui, du fait de la perte de l'allocation peuvent entrer dans une relation de dépendance au nouveau conjoint plus beau but plus globalement ces débats ne sont pas si éloignés de ce que nous avons pu avoir, il y a quelques semaines autour de la dope l'allocation adulte handicapé dans les 2 situations, un seul et même objectif doit nous guider, permettre l'indépendance face à une difficulté de la vie et faire en sorte qu'aucune considération financière puisse influencer des choix de vie, s'y ajoutent, dans le cadre de l'ASM, l'intérêt supérieur de l'enfant aussi cette suspension du versement de l'ASM en cas de retour à une vie de couple pour l'un des parents est d'autant plus incompréhensible qu'il n'y a pas de conditions d'isolement pour le versement de la pension alimentaire, comment expliquer cette différence entre 2 types de familles monoparentales, au-delà de l'incompréhension, ce statu quo viennent nourrir la fraude et à ce titre, je regrette que nous, la majorité sénatoriale ne donne pas davantage d'écho à cette proposition de loi si la réforme des politiques sociales et nécessairement continue : je souhaite que l'élection présidentielle présidentielle viennent remettre au débat, ces sujets comme celui de l'allocation adulte handicapé ou encore le non-recours aux aides sociales, ou ce sont près de 10 milliards qui ne pourrait être mobilisés en plus chaque année, si je suis favorable à cette proposition de loi, certaines d'entre nous sont plus partagés, souhaitant notamment une remise à plat de cette allocation et des objectifs qui lui sont affectés ou encore une réforme plus globale et de nos piles politique sociale aussi, et vous l'aurez compris les membres du groupe RDSE, dans leur grande majorité voteront cette proposition de loi je vous remets. Merci, la parole est à Madame Annie. Le verrou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes chers collègues.

Madame la présidente, monsieur le ministre madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui représente une avancée majeure pour les parents isolés, actuellement, l'allocation de soutien familial a pour objectif d'aider à l'éducation d'enfants privés du soutien d'au moins un des parents, lorsque ce dernier défaillants ou absents. Cette allocation vise en priorité les femmes monoparentales les plus vulnérables surexposés à la pauvreté, l'allocation de soutien familial et versée à 807000 familles et bénéficie à 3 millions d'enfants actuellement, dès lors que le parent se met en couple le versement de l'ASF supprimé. La présente proposition de loi de ma collègue Laurence Rossignol, dont on connaît la détermination à défendre l'intérêt des enfants et je salue ici son travail incessant, cette proposition vise à supprimer cette condition d'isolement pour bénéficier de l'ASF, afin de permettre à des parents en famille recomposée de recevoir cette allocation, en effet, ce mécanisme de suspension repose sur l'hypothèse contestable et moralement inacceptable que le nouveau partenaire de vie contribuent automatiquement à l'éducation des enfants, l'obligation alimentaire est alors déporté sur une personne qui n'a aucun lien de parenté avec l'enfant d'ailleurs dans la plupart des situations, cette hypothèse ne reposent sur aucune réalité concrète, mais certains parents isolés sont contraints de faire un choix : soit se remettre en couple et renoncer à l'allocation, c'est-à-dire se retrouver avec des difficultés financières encore plus prégnante ou renoncer à une nouvelle vie de couple c'est inacceptable l'octroi de cette allocation ne doit pas être lié à un critère de conjugalité en France aujourd'hui, près de 2 millions de de familles sont monoparentales, soit une famille sur quatre ces familles sont 2 fois plus touchées par le chômage et la précarité, les familles monoparentales sont constituées à 85 % de mères et de leurs enfants, leur nombre est en forte augmentation du fait de la hausse de séparation, d'après l'Insee, 12,5 % des femmes tombent dans la pauvreté après une séparation. Cette situation nécessiterait la reconnaissance d'un statut de mono-par permettant de bénéficier d'un accompagnement dans la vitre la vie quotidienne, proposition qui trouvera sa place dans la campagne présidentielle derrière la qualification de familles monoparentales se cache une réalité quotidienne très compliqué ces mères isolées doivent jongler entre l'éducation des enfants, une forte charge mentale, l'organisation de la prise en charge de chaque enfant et lorsque c'est possible, une activité professionnelle qui est parfois difficile à assumer, elle doit faire de nombreux sacrifices qui ont inévitablement un impact sur l'activité professionnelle, emploi ou formation mais également sur leur vie personnelle, les empêchant de disposer de moments de répit, la constitution de réseaux d'entraide est rendue difficile par cette faible disponibilité pour nombre de mères monoparentales se mettre en couple représente une opportunité de soulager la charge familiale qui pèse uniquement sur elle, celles qui ne peuvent pas se passer de l'ASF pour leur survie matérielle sont contraintes de rester célibataire avec un niveau de vie médian avoisinant 1180 euros mensuels bien en-deçà du revenu médian, la moitié de ces familles vivraient avec ce faible niveau de revenus en 2020, 24000 par an aurait perdu le bénéfice de cette allocation, alors qu'ils ont choisi de se remettre en couple. La perte de cette allocation peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis de leurs nouveaux partenaires le ciblage de l'ASF sur les seuls parents isolé constitue donc une double peine pour ces personnes. Le bénéfice de l'ASS au seul parent isolé déclenche une forme de trappe à l'isolement, ça a déjà été dit qui constitue une entrave à la remise en couple, par ailleurs, en raison de la complexité des conditions d'octroi l'ASF est concernée par un important phénomène de non-recours à cela s'ajoute un non-recours volontaire, les maires concernés préfèrent renoncer à cette allocation et éviter d'engager un litige avec leur ancien conjoint défaillant ainsi près d'un parent isolé sur 2 seraient éligibles à l'ISF, mais ne la réclamerait pas, vous l'avez d'ailleurs repris, Monsieur le Ministre, cette condition d'isolement constitue un obstacle supplémentaire à la à l'octroi de cette allocation déjà difficilement accessibles aux personnes concernées. En supprimant cette condition, ce texte propose une réponse concrète et une incohérence des modalités d'attribution de l'ASF. Une réponse concrète à l'incohérence des modalités d'attribution de l'ASF, l'ASM doit être considérée comme une allocation pour le parent qui assume seule l'éducation de ses parents, indépendamment de sa situation de couple souvent non stabilisée, le maintien de l'allocation aux parents éligible à des. Prudemment, de la condition d'isolement est une mesure de justice sociale pour les familles concernées, leur évitant de basculer dans la précarité, les familles monoparentales étant principalement constitués par des maires, cette mesure de bon sens permet à ces femmes de conserver leur indépendance économique vis-à-vis de leurs nouveaux partenaires ainsi à l'issue de la discussion, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera favorablement et sans réserve pour cette proposition de loi qui aidera à la subsistance des personnes en situation de monoparentalité et rendra moins difficile, la situation de précarité que vivent la moitié d'entre elles. Merci, merci, cher collègue, la parole est à monsieur Martin lévrier. Pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 4 minutes.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, l'allocation de soutien familial, anciennement connu sous le nom d'allocation parent isolé, est versée pour soutenir les parents qui élèvent seules leur enfant 815000 foyers français ont ont bénéficié, pour un coût total d'1,60079 milliards d'euros, cette prestation est conditionnée à l'isolement du parent lorsque le parent bénéficiaire se remettent en couple, il perd la prestation, mes chers collègues, en 2020 la France comptait 2 millions de familles monoparentales, soit 24,7 % de l'ensemble des familles, soit 2 fois plus qu'en 1990 l'augmentation de la proportion de ces familles et des familles recomposées, constitue un fait social auquel les dispositifs sociaux, fiscaux ont dû s'adapter de plus, les chiffres de l'Insee ne prenne ne prête pas à controverse dans un tiers des familles monoparentales, le parent avec lequel il réside la plupart du temps n'a pas d'emploi. Cette réalité a des réponses fortes, soit par le biais de prestations ciblant spécifiquement les parents isolés, soit en prévoyant une majoration de accordés, soit au travers de plafond de ressources pour ces publics, c'est le cas pour le RSA, mais aussi pour la majoration du plafond du complément de mode de garde par exemple. Ces majorations spécifiques perdent leur effet dès lors que le parent isolé, soumis à nouveau un un nouveau partenaire de vie. Le texte déposé par Madame Laurence Rossignol que nous examinons aujourd'hui vise dans son article 1er à supprimer le conditionnement du célibat pour obtenir l'allocation de soutien familial. Part du principe que le nouveau partenaire de vie n'a aucune obligation de s'impliquer dans les dépenses liées à la prise en charge des enfants de la personne avec laquelle il entend s'unir le second article de la PPL vise quant à lui, a demandé au gouvernement un rapport sur la diversité des situations familiales et leur prise en compte par la fiscalité, si ce texte est louable dans ses intentions, bien évidemment, il soulève un certain nombre de réserves pour 3 raisons essentielles. Premièrement, ces nouvelles dispositions, risquerait de remettre en cause l'application des autres, ce dispositif précités qui sont mises en oeuvre au profit des parents isolés. Deuxièmement, une telle mesure risquerait de n'avoir qu'un faible impact sur les publics les plus précaires que notre politique familiale entend cibler en priorité, force est de constater que les enfants qui grandissent avec un couple au sein d'une famille recomposée ou non, ont un meilleur niveau de vie que ceux qui évolue au sein d'une famille monoparentale, troisièmement, alors que la France consacre un pays, un pourcentage de son PIB, plus important que la moyenne de l'Union européenne, celle de l'OCDE, il eut été indispensable que le coût financier de cette PPL soient chiffrées, par ailleurs, nous savons que 85 % des foyers monoparentaux sont constituées de femmes, il est d'évidence que cet appel, cherchent à améliorer leur indépendance économique. Ce sujet a régulièrement été la priorité du gouvernement, par exemple, nous avons voté pour les familles éligibles à l'ASF, la possibilité de bénéficier d'une facilité dans la garde d'enfants pour les parents, engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, nous croyons profondément qu'on accompagnant la prise en charge des enfants et l'insertion du sans emploi, nous aidons ces familles encore nous avons réformé les pensions alimentaires, enfin, n'oublions pas que le taux de non-recours à l'ASF est extrêmement élevé et je pense que c'est sur ce point que nous devons concentrer toute notre attention et nos intentions. Pour ces raisons, et malgré le fait que nous partagions bien évidemment l'objectif affiché notre groupe votera en majorité contre cette PPL je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Joël Guerriau pour le groupe, les indépendants, République et Thierry victoire et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre. Cette PPL s'inscrit dans la volonté du bien-être des enfants puisqu'elle propose de revoir d'une des conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, cette allocation n'est perçu que dans des cas particuliers respecte plusieurs modalités dont celle d'être ni marié ni liés par un Pacs, ni même d'être en concubinage, l'allocation de soutien familial a évolué au cours de son histoire, mais nous devons garder en tête que le destinataire reste et doit demeurer l'enfant, nous parlons de son, d'éducation et de son avenir et je salue la réflexion qu'il y a autour de ce texte, ainsi que l'engagement qui suscite à la qualité de nos débats, nous comprenons les difficultés auxquelles font face les familles percevant cette allocation, les familles monoparentales sont souvent confrontés à des préoccupations particulières et persistante, nous entendons aussi des arguments qui ont été donnés la dépendance économique vis-à-vis du nouveau conjoint la situation familiale de ce dernier ou encore sa volonté ou non d'application dans l'éducation de l'enfant, nous comprenons donc bien la volonté qui est mise dans ce texte, mais ce qui est proposé ne répond pas à toutes nos interrogations, j'évoquerai seulement 2 points qui ont été soulevées en commission le 1er et le fait d'assumer la recomposition de la famille en prenant en compte l'éducation à la charge des enfants, cela me paraît essentiel dans le cas de mariage ou de Pacs d'autant plus que certains ont avancé le fait que le parent qui a en charge l'enfant pourrait préférer rester seul, évoquant des problèmes de fiscalité, il est d'ailleurs regrettable que des considérations fiscales prévalent sur la recomposition d'une famille pour autant dans le cas du mariage, du Pacs, les nouveaux conjoints et les enfants, même lors de la garde partagée font partie du même foyer fiscal et, de fait, bénéficie d'un quotient familial pouvant réduire le niveau d'imposition ainsi, il serait nécessaire, finalement, d'approfondir tous ces mécanismes pour prendre en considération la différence entre toutes les situations de fait et de droit cette-là n'amène m'amène donc un second point une réforme en profondeur du système des allocations, plutôt que de petites modifications, aussi importantes soient-elles, cette réforme globale ne pourra se faire que si nous évoluons et nous faisons évoluer le système actuel dans son ensemble, ces faiblesses comme s'forces devront donc être clairement identifiés : l'une de ses faiblesses et le contrôle du bon fonctionnement du système malheureusement les fraudes aux allocations familiales sont très nombreuses et concernent les différents types d'allocation, notamment les fraudes à la résidence ou à l'isolement et là il faut bien sûr lutter contre ce phénomène, rappelons que d'après un rapport de la Cour des comptes, de septembre 2020 les fraudes sociales détectées se situe autour d'un milliard d'euros au sujet des fraudes non détectés, le chiffre serait compris entre 14 et 45 milliards d'euros, ce qui bien sûr est tout à fait énorme et avant d'élargir l'accès aux allocations, ne faudrait-il pas, au préalable, récupérer ce qui est injustement perçues par des fraudeurs, maître de l'Ordre dans le contrôle qui est fait et se lancer dans une réforme profonde du système et bien plus que nécessaire, cela nous permettra surtout de pouvoir concentrer nos efforts en faveur de nos concitoyens qui en ont le plus besoin et au 1er desquels les familles monoparentales, si nous partageons donc l'idée générale dégagée par cette PPL nous préférerions qu'une réflexion plus affronte plus approfondie, nous permettent d'engager une réforme de plus grande ampleur et c'est pourquoi le groupe les indépendants s'abstiendra. Si cher collègue, la parole est à madame Chantal de scènes qui ne va pas tomber dans les escaliers, mais va vous voulez. C'est le temps pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes chers collègues. collègues. Présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour examiner la proposition de loi visant à maintenir le versement de l'allocation de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses du parent bénéficiaire, créé par la loi du 22 décembre 1984 l'ASF est versée par la branche famille, c'est une prestation familiale qui peut être versée aux personnes à la mer, seule ou à toute autre personne. Ayant recueilli un enfant et en ayant la charge effective et permanente,

l'allocation de soutien familial et versées sans conditions de ressources, son montant s'élève à 116 euros par mois et par enfant à charge, elle est attribuée par les caisses d'allocations familiales ou mutualité sociale agricole, l'ASF également être attribué pour compléter une pension alimentaire dont le montant est inférieur à 116 euros ou être versées à titre d'avance quand celle-ci n'est pas réglée par l'autre parent, dans ce cas, la CAF engage une procédure de recouvrement auprès de ce dernier pour la récupérer cette prestation est accordée aux parents ayant la charge de l'enfant, sous réserve de son isolement et cesse donc d'être versés si le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation Revit en couples ou si les enfants sont en garde alternée, il s'agit d'une prestation destinée à l'enfant, selon l'Insee, on compte en France plus de 2 millions de familles monoparentales, soit environ une famille sur quatre les familles monoparentales sont particulièrement exposés aux situations de précarité en raison de ressources financières moindres ou d'un risque de chômage, plus élevée que celle formée d'un couple avec enfants, c'est pourquoi le système français prend déjà en compte la monoparentalité par de nombreux dispositifs ainsi les parents isolés peuvent aussi prétendre au système de double plafond favorable mises en place pour le complément familial à la modulation à la hausse du montant de certaines prestations légales à l'allongement de la durée du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui peut être allouée pendant 6 mois supplémentaires en cas de monoparentalité les parents isolés peuvent aussi bénéficier de l'aide à la garde d'enfants pour parent isolé afin de faire garder un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans lorsqu'ils retrouvent un emploi à temps il bénéficie aussi d'une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt qui est également accordée aux parents seuls sans personne à charge qui a élevé seule ses enfants au moins 5 ans, cette proposition de loi va plus loin et demande le maintien du versement de l'allocation de soutien familial en cas de nouvelles relations amoureuses et parents bénéficiaires je pose donc la question de savoir si tous les dispositifs destinés aux parents isolés devront à terme être aussi maintenu en cas de nouvelles relations amoureuses du parent bénéficiaire, ça n'a pas de sens, vise à apporter un soutien ciblé aux monuments aux familles monoparentales, en raison de la situation particulièrement précaire dans laquelle elle se trouve, le maintien de cette allocation n'a pas lieu d'être, à partir du moment où le parent isolé se remet en couple, la suspension du versement de l'ASF repose en effet sur le postulat que le nouveau conjoint participent à l'entretien de l'enfant, le vrai problème est que depuis le quinquennat de François Hollande, le détricotage de notre politique familiale et continue les mesures d'économies mises en Oeuvres par les gouvernements successifs ont impacté directement le budget des familles qu'il s'agisse de la modulation des allocations familiales, de la suppression du complément de libre choix d'activité majoré de la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, il serait plus opportun de proposer des mesures afin d'apporter des réponses adaptées aux inquiétudes des familles monoparentales, quant à la conciliation de leur vie professionnelle et familiale, il faut développer, entre autres, des solutions d'accueil pour les jeunes enfants, supprimer les conditions de ressources du complément mode de garde, permettre aux parents isolés et aux couples de travailler sans encourir un reste à charge dissuasif pour la garde à domicile, comme pour les crèches et les assistantes maternelles, le mouvement doit être inversée autour d'un nouvel universalisme, c'est toutes les familles qui doivent être soutenus, la famille, la politique familiale constitue un investissement pour l'avenir, qui ne peut se contenter d'aménagement à la marge, notre politique familiale, a besoin d'un vrai sursaut pour conclure, je pense qu'il faut le courage de remettre à plat toute la politique familiale et privilégier le principe d'universalité, plutôt que des mains d'aménager à la marge des allocations spécifiques. Pour toutes ces raisons, le groupe Les République là il ne soutiendra pas cette proposition de loi. Même si cher collègue, la parole est à Madame Raymond. Forcément, pour le groupe écologiste solidarité et territoires et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, si les vulnérabilités. Femmes hommes puis souvent leur source dans la structure normative qui cadrent les relations, c'est la séparation conjugale qui révèle brutalement les inégalités creusées. Durant toute la vie de couple. Dans leur livre le genre du capital ou comment la famille reproduit des inégalités, les chercheuses baissière et que et Gola qui souligne que les effets différenciés d'une séparation résulte de stratégies économiques et qui ont eu lieu dans la la conséquence d'une répartition inégale des rôles économique dans le couple, temps des stratégies de dépenses que de la division genre et du travail professionnel et du travail domestique gratuit, explique que le prix de la rupture est encore aujourd'hui chèrement payée par les femmes, en effet, une séparation, conduit à une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes, contre seulement 2 5 % pour les autres, ces inégalités vont perdurer puisque presque 84 % donc presque 84 % des cas, les familles monoparentales sont constitués de mer et 40 % des enfants de ces familles. Sont pauvres, ces mères sont davantage au chômage occupent plus souvent des postes précarisés suite des carrières plus heurtées. Aussi venant compenser parfois la faiblesse de certaines pensions alimentaires, les parents bénéficiaires de la le. Question du est ce que vous pouvez vous mettent au milieu des 2 micros Sylvain Bourget merci beaucoup. Aussi venant compenser donc parfois la faiblesse de certaines pensions alimentaires, les parents bénéficiaires de l'allocation de soutien familial à partir pour plus de 70 % au 20 % des ménages les plus pauvres, la suppression de cette allocation dans le cas de la reconstitution d'une nouvelle famille repose donc sur le postulat que celle-ci est automatiquement créatrice de nouvelles solidarités qui rendrait caduque. Prestation mais en réalité, la recomposition d'un coupe-n'efface pas pour autant la situation personnelle vulnérable d'une majorité de ses parents et de plus on ne sort pas de la précarité en se mettant simplement en Coupe, surtout si l'autre est aussi précaire, surtout qu'on perd cette prestation lors d'une remise en coupe prestation pour soutenir les frais d'éducation de l'enfant, c'est une marge d'autonomie financière qu'on perd et une dépendance économique et symbolique qui se crée, car ce nouvel espace de solidarité ne génère pas pour autant pour le nouveau partenaire des obligations envers l'enfant comme celle qu'aurait eu le parent dont il est privé la prestation doit demeurer attaché à la situation inchangée de l'enfant, là réside son sens profond, enfin on ne peut exclure la des incitations à s'engager pour les plus fragiles du fait de la baisse immédiate de revenus accompagnant la perte de cette prestation de soutien essentiel à ces niveaux de revenus en conséquence le maintien du versement de cette allocation, indépendamment de la situation affectif du parent qui en assure l'éducation permette de stabiliser la situation et de s'engager dans une nouvelle relation sans impact collatéral sur une allocation dont l'objet est la fonction n'ont aucunement disparus, le texte de loi proposée tient compte de l'augmentation des familles recomposées et adapte donc le droit aux évolutions sociétales pour le groupe écologiste s'attaquer ainsi aux trappes à pauvreté ou à l'isolement comme aux inégalités de genre qui les traversent reste une priorité, une urgence, aussi nous voterons cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole. Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier nos collègues socialistes et particulièrement Laurence Rossignol et Michelle Meunier, d'avoir mis en lumière cette problématique assez peu connu et qui nécessite en effet un changement car en se plongeant dans le dispositif de l'allocation de soutien familial et de son ancêtre, l'allocation d'orphelins, on constate que la législation n'a que peu suivi l'évolution de la société et la composition des ménages cette prestation apparaît aujourd'hui anachronique, fondée sur un critère de célibat fixé par la loi du 23 décembre 1970 cette année 1970 est aussi l'année où est instauré l'autorité parentale conjointe supprimant la notion de chef de famille du code civil, c'est aussi l'année du 5ème anniversaire de la loi autorisant les femmes à travailler et à ouvrir un compte en banque sans le consentement et l'autorisation préalable de leur mari, et il faudra encore attendent 23 ans, pour que s'affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants quelle que soit la situation des parents si je fais ces quelques rappels historiques, c'est pour tenter de mieux comprendre l'esprit du législateur au moment de créer ce dispositif est de mesurer son idée inadaptation en 2022, en réalité, ce critère de célibat est inopérant à plus d'un titre, premièrement, si le Pacs et le mariage sont des modalités d'union comportant une obligation de solidarité entre les conjoints, ce n'est pas le cas par exemple du coup nage l'automaticité fait entre relations amoureuses officialisé et partage financier des charges n'a donc pas de réalités tangibles, deuxièmement, et malgré l'obligation de solidarité que j'évoquais précédemment, il est impossible d'établir que chaque couple marié ou pacsé partage bien les charges financières, troisièmement, le dispositif est facilement contournable, il suffit aux parents célibataires, engagés dans une nouvelle relation de ne pas officialiser cette relation, or cette décision, a des conséquences non négligeables sur le court, moyen et long terme en matière de fiscalité ou encore de succession et ce au détriment des parents célibataires ensuite secrétaire maintient l'ambiguïté sur le destinataire final de l'allocation est l'enfant ou le parent célibataire pour nous, c'est bien l'enfant qui doit en être le bénéficiaire et fonder son attribution en fonction du statut matrimonial de ses parents est une aberration et créent une rupture d'égalité entre les enfants, enfin, ce critère est profondément injuste puisqu'il demande aux parents célibataires soit d'abandonner leur allocation de soutien familial et de se mettre en quelque sorte sous la coupe financière de nouveau conjoint soit de renoncer à une nouvelle vie de couple pour conserver le bénéfice de cette prestation, c'est d'autant plus problématique qu'on parle ici d'un dispositif qui touchent les familles les plus fragiles économiquement et socialement, si l'on regarde les chiffres de l'Insee de septembre dernier, les familles monoparentales sont celles où on trouve le plus de familles dans des logements surpeuplés, où le taux de pauvreté des enfants est largement supérieur au taux de pauvreté moyen pour la même classe d'âge, et où le taux de non-emploi des parents est supérieur au sein même de ces familles, les mères qui représentent 82 % de l'ensemble des familles parental sont plus mal lotis que les pères, elles vivent avec plus d'enfants en moyenne, sont plus souvent en situation de pauvreté et moins souvent en situation d'emploi lorsqu'elles travaillent, elles sont plus souvent en situation précaire ou dans des emplois les moins rémunérateurs dans ce contexte, l'ASF est une ressource essentielle pour qu'elle puisse espérer s'en sortir financièrement, ils n'ont, il n'est donc pas acceptable qu'un critère aussi injuste et incohérent que le célibat présumés viennent remettre en question cette prestation, c'est pourquoi notre groupe, le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste votera cette proposition de loi avec enthousiasme. Merci, cher collègue, la discute. Jean générale est Close, la commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi. Initial Madame Madame la Présidente Rossignol.

un soutien bienveillant par l'abstention ou le vote à ce texte et qui ont relevé que cette proposition de loi Elvis quand même à mettre en exergue, une situation qui est très incohérente et en fin de compte, herbe qu'emprunte d'un moralisme très archaïque, ce que dit le texte que je propose de supprimer avec mes collègues, c'est lorsque le père ou la mère titulaires de l'allocation se marient conclu un pacte civil, ça ce sont des situations juridiques ou vit en concubinage, l'allocation est supprimé, or je me suis replongée dans dont les les la CAF identifie des situation de concubinage qui sont par définition des situations dans lesquelles il n'y a pas de d'encadrement juridique la situation de concubinage, elle se défini par des une communauté d'intérêts sur le plan affectif la charge matérielle et affective des enfants qui n'est pas systématique, loin de là, malheureusement, peut-être dans la remise en couple et qui se défini défini par un contrôle de la notoriété de la vie commune établie à partir d'enquêtes de voisinage auprès des services de police et de gendarmerie, il y a là quand même, de quelque chose qui est assez étrange, si cette même personne retourne habiter chez ses parents où elle bénéficiera d'un soutien matériel, elle paiera une sa contribution aux charges locatives sera moins grande, elle pourra aussi bénéficier d'un soutien affectif, elle continuera paix de percevoir l'allocation de soutien familial si elle vit avec une amie. à moins d'une enquête de voisinage très poussée pour aller voir la nature de sa relation avec son ami, elle continuera de bénéficier de l'allocation de soutien familial, mais si elle vit avec un homme. Elle ne pourra plus bénéficier de l'allocation de soutien familial parce que il y aura le contrôle de notoriété de la vie commune et une présomption de relation affective, je voudrais juste quand même que vous êtes vous appréhende yé à quel point. Cette ce 2ème alinéa de cet article du code de la sécurité sociale et anachronique et moraliste, merci. Sur l'article 1er j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, voilà, nous avons une niche la dernière niche de notre session avant la pause et manifestement l'intérêt pour les chômeurs de longue durée ou pour les situations évoquées par Madame Rossignol ne mobilise pas totalement la majorité sénatoriale ce qui vous amène à multiplier systématiquement le scrutin public je regrette cela c'est pas une bonne image pour le fonctionnement normal de notre démocratie et de notre institution de la Haute Assemblée, je vais vous le dire par ce rappel au règlement.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Alors voici le résultat du scrutin numéro 114 sur l'article 1 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs au groupes politique et notifié à la présidence, nombre de votants 340 Nombre de suffrages exprimés 268 pour l'adoption 103 contre 165, le Sénat n'a pas adopté alors, mes chers collègues, je vais mettre aux voix l'article 2 je vous rappelle que si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les 2 articles qui la composent, aurait été supprimés, il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur l'ensemble, est ce que quelqu'un demande la parole pour expliquer son vote. on a déjà eu la discussion, il y a peu de temps à propos de la la PPL. Proposé par notre collègue sur la politique familiale et je pense qu'on ressent tous, peut-être avec des angles de vue différents le besoin d'une vraie réflexion collective du pays sur la politique familiale, ces enjeux et, surtout, c'est son objet et je pense que je crois que c'est Élisabeth Doineau qui l'a dit tout à l'heure, une des évolutions principal de la politique familiale, c'est qu'elle est désormais centrée sur l'enfant, et ça, beaucoup de conséquences sur l'approche de la politique familiale et pourquoi nous demandons ce rapport parce que la politique familiale, c'est effectivement les prestations familiales versée par les CAF, mais c'est aussi des politiques fiscales en particulier j'ai évoqué tout à l'heure la question du de par le plus souvent, les maires des pensions alimentaires qu'elles perçoivent alors que le père lui déduit ses pensions alimentaires de ses revenus imposables : nous aimerions avoir un jour des éléments de des services fiscaux sur l'impact d'une évolution sur ce sujet et puis les questions de déconjugalisation d'autonomie fiscale sont des questions qui sont posées et je dis en particulier mes collègues de la droite du sénat qui ont porté la déconjugalisation de l'AAH que cette réflexion ne peut pas s'arrêter à la question de l'allocation adulte handicapé, c'est l'ensemble de nos politiques sociales et familiales, qui doit être non pas totalement revu, mais au moins, pour lesquels nous devons avoir les éléments et donc peut-être le Sénat exceptionnellement par cohérence avec ses propres propositions de loi pourrait voter cette demande de rapport. Merci monsieur Bush. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, être majoritaire dans une assemblée, c'est un honneur, mais cela confère quelques obligations et parmi ces obligations s'astreindre à une présence minimale et ne pas recourir systématiquement aux artifices de procédures et au scrutin public comme nous avons assisté ce soir depuis que je siège au Sénat, à chaque fois qu'un groupe politique de la majorité ou de la minorité a déposer ou de l'opposition a déposé des propositions de loi dans une niche parlementaire, il y a des règles de courtoisie républicaine qui font que chaque groupe politique s'astreint assurent une présence et à nourrir le débat, on ne peut pas venir ici ce soir, nous jurer la main sur le coeur que la précarité des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, les chômeurs de longue durée que la précarité des familles monoparentales et quelque chose de grave et de sérieux et finalement venir systématiquement empêché le débat comme nous y avait assisté ce soir, je le regrette vraiment et sincèrement. Merci, Monsieur le Ministre. Miniaturisé, il y a des prises de parole non, simplement, de 2 choses, en en réponse à l'intervention notamment de Laurence Rossignol et à cet article de dire que cet article 2 est en quelque sorte, satisfait et je rejoins mais je rejoins sur le fond.

des dépenses en matière de politique familiale, puisque effectivement il y a une dimension sociale, fiscale très conséquente dans notre dans notre politique familiale et non les inspections ont dit qu'elle ne correspondait pas plus forcément à la réalité des familles contemporaines et il y a probablement un grand soir social ou fiscal de la politique familiale à faire dans notre pays, peut-être qu'il arrivera dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, 2 autres rapports commandés au FC cette fois-ci, d'une part, un 1er sur le bilan des 20 dernières années des politiques familiales, et un second panorama que j'ai demandé, moi je sais faire de dresser sur les sur le le les familles contemporaines en insistant en se focalisant sur quatre non pas un modèle de manière famille contemporaine que sont les familles monoparentales, les familles homoparentales les familles nombreuses qui reste, qui reste une composante importante des familles d'aujourd'hui et puis les familles recomposées, évidemment je l'ai évoqué dans mon intervention, je pense que la question de la séparation de la recomposition les droits envers envers les beaux enfants reste encore des champs à à explorer dans notre palette Typhaine et puis second point donc voilà votre article 2 est satisfait, quelle que soit on aime la la rapporteure et je vous invite donc à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, comme nous y a invités Laurence Rossignol a plongé dans ces 3 rapports, vous y trouverez beaucoup de matière à à réflexion et vous dire par ailleurs

depuis 20 à 30 ans avaient tendance à tourner justement autour des seules questions fiscales ou se ou faut-il bouger le quotient familial : Faut-il bouger le niveau des allocations, les débats se sont souvent concentrées limitées à ce genre de de considérations, ça ne veut pas dire que la dimension monétaire n'est pas importante évidemment dans la politique familiale, la question de la redistribution horizontale dans demeure pas une composante toujours pertinentes pour autant nous assumons d'une part que la petite familiale est une politique sociale de redistribution également verticale s'était présenté le plan de lutte, de prévention et de lutte contre la saisie de la contre la pauvreté ou l'enfant, effectivement, était au coeur de sa stratégie de lutte contre la pauvreté et puis par ailleurs, nous pensons qu'il ne faut pas parler uniquement de l'universalité des des allocations familiales, qui est un peu un devenu un peu un totem, en réalité, on peut se le dire, mais qu'il fallait vers une universalité des services de passer effectivement une politique familiale vers une politique d'accompagnement à la parentalité, où l'enfant est au coeur de notre de notre politique, et c'est vrai qu'avoir l'enfant comme prisme de la politique familiale, nous permet de redécouvrir totalement ce Champ, c'est ce que nous essayons de mettre en oeuvre depuis 3 ans, notamment avec la politique autour des 1000 premiers jours de l'enfant, mais c'est un chant qui reste encore largement à explorer, voilà ce que je voulais partager et j'en profite pour conclure je ne demanderai pas la parole pour vous remercier toutes et tous, vous qui êtes là ce soir et puis tous ceux qui ne sont pas là pour les 3 ans partagé en votre compagnie qui ont été fort riche passionnants, intéressants intense et puis remercie surtout fin également tout le personnel du Sénat les huissiers, les administrateurs de toutes les personnes qui concourent à ce que nous puissions débattre et à ce que la démocratie reste vivace dans notre pays, merci à tous. Merci monsieur le ministre. Alors, je vais mettre aux voix l'article 2 pour lequel j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Voici le résultat du scrutin numéro 115 sur l'article numéro 2 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 340 Nombre de suffrages exprimés 268 pour l'adoption 103 contre 165, le Sénat n'a pas adopté les articles de la proposition de loi ont été successivement supprimé par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte en conséquence, la proposition de loi n'est pas adopté, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance jeudi 24 février à 10 heures 30 pour le débat, à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes, la seule séance est levée.